Monsieur le président,

La séance est reprise.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Président de la République s'est exprimé hier pour présenter à la Nation les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de covid-19 qu'il convient désormais de mettre en place. Une fois encore, vous le savez, la France doit affronter les assauts de cette crise sanitaire, une crise sanitaire qui dure depuis très longtemps, avec un virus qui mute et évolue de manière inquiétante. Alors, une fois encore, nous devons faire face. Nous devons prendre en toute connaissance de cause les décisions que la situation impose. La gravité de cette troisième vague- d'une certaine façon, c'est une nouvelle épidémie l'impact de ces décisions sur nos concitoyens qui font face courageusement, et depuis des mois, à cette pandémie mondiale, tout cela exigeait que les représentants de la Nation puissent en débattre et s'exprimer par un vote solennel dans le cadre fixé par l'article 50-1 de la Constitution. Je suis venu vous dire cet après-midi que ces mesures nouvelles nous apparaissent maintenant indispensables pour protéger la vie et la santé de beaucoup de nos concitoyens, particulièrement les plus fragiles. Elles sont indispensables ... Sauf pour les Anglais ! ... pour permettre à notre pays de franchir ce que nous espérons toutes et tous être une dernière étape, dans la perspective du déploiement massif de la vaccination et donc d'un retour à une vie normale. La troisième vague déferle et frappe durement. L'épidémie s'emballe depuis la mi-mars : en deux semaines, le nombre de cas a augmenté de 55 % pour s'élever aujourd'hui à environ 38 000 par jour. L'épidémie progresse vite et partout. Cette forte accélération est, chacun le sait, le résultat de la progression du variant apparu en fin d'année dernière en Grande-Bretagne. Nous savions qu'il était plus contagieux. De récents travaux scientifiques prouvent qu'il est aussi plus dangereux. Comme je le constate à chacune de mes visites dans des établissements de santé, le virus frappe des patients plus jeunes jeunes et, en plus grande proportion, des patients sans facteur de risque lié à des comorbidités. Bien évidemment, ce phénomène n'est pas propre à la France France : depuis une quinzaine de jours, le nombre de cas quotidiens a triplé en Allemagne et il a augmenté de 70 % en Belgique et de 40 % aux Pays-Bas. Cette virulence accrue de l'épidémie est particulièrement préoccupante, car elle survient à un moment où notre système de santé est déjà mis à lourde contribution, et ce depuis longtemps. Avec plus de 5 000 malades de la covid-19 hospitalisés en réanimation, c'est certes moins que le pic de la première vague, mais celui de la deuxième vague est désormais dépassé. Face à ce nouveau virus, nous avons rapidement réagi, en prenant ces derniers mois et semaines plusieurs mesures fortes maintien depuis fin octobre de la fermeture de nombre d'activités et établissements recevant du public, couvre-feu national depuis la mi-décembre, mesures renforcées dans près de 20 départements couvrant près d'un tiers de la population, et ce depuis le 20 mars dernier. Nous l'avons fait en tenant le plus grand compte des différences de situation territoriale- étaient particulièrement perceptibles en début de vague épidémique. Si j'insiste ici, devant la Haute Assemblée, sur la territorialisation des mesures que nous avons prises, c'est parce que je sais à quel point les membres du Sénat étaient, tout comme moi, attachés à une adaptation de notre politique sanitaire aux réalités du terrain. La stratégie de réponse territorialisée que nous avons utilisée depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui était la bonne, car l'épidémie frappait alors nos territoires de manière très hétérogène ; il n'y avait pas de raison d'appliquer un durcissement des mesures dans les territoires où le virus circulait très peu. Mais, aujourd'hui, le variant britannique poursuit son accélération dans de telles conditions que nous devons nous aussi accélérer, c'est-à-dire prendre des mesures renforcées, de façon à briser la spirale épidémique enclenchée depuis quelques semaines. variant accélère malheureusement sur l'ensemble du territoire métropolitain. Depuis une dizaine de jours, sur 96 départements, 92 connaissent une accélération de la circulation virale avec des rythmes parfois spectaculaires supérieure à 20 % sur une semaine dans la moitié des départements et de plus de 40 % dans une vingtaine d'entre eux- c'est par exemple le cas du département des Pyrénées-Orientales, où le taux d'incidence a progressé de 73 % en sept jours. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, sous l'autorité du Président de la République, d'étendre à l'ensemble du territoire métropolitain les mesures qui s'appliquaient déjà dans les 19 départements les plus touchés par l'épidémie. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur samedi soir à 19 heures pour être pleinement applicables le dimanche 4 avril, et ce jusqu'au 3 mai, soit pour une durée de quatre semaines. Face à la situation actuelle, il nous faut agir fortement à l'échelle nationale, selon les mêmes règles et les mêmes calendriers pour tous. En prenant une mesure nationale, nous souhaitons aussi préserver l'offre hospitalière des régions moins durement touchées, qui pourraient fournir des capacités de repli pour les régions davantage en tension. Il nous faut cependant faire une exception pour les collectivités et départements d'outre-mer, dont la situation sanitaire n'est évidemment pas comparable à celle de la métropole, ni même du reste d'un territoire à l'autre, compte tenu de leur éloignement géographique. continueront donc à observer des règles spécifiques et adaptées aux évolutions épidémiques propres à chacun d'entre eux. Comme l'a indiqué hier le Président de la République, les règles qui s'appliqueront à compter de samedi soir au territoire métropolitain seront identiques à celles qui ont été mises en place depuis le 20 mars dernier dans les 19 départements soumis à des mesures renforcées. Le couvre-feu sera maintenu à 19 heures. L'ouverture et la fermeture des commerces obéiront aux mêmes critères et conditions. Le télétravail sera systématisé quatre jours par semaine au minimum pour tous les emplois publics et privés, quand cela est possible. Les motifs de sortie et de déplacement seront encadrés selon les mêmes termes : il restera possible de se déplacer, de se promener, de faire du sport, sans limitation de durée et dans un rayon de dix kilomètres autour de chez soi. En revanche, les rassemblements ou regroupements de plus de six personnes resteront interdits. Enfin, une attestation précisant le motif du déplacement sera exigée au-delà des dix et, après la fin du prochain week-end prolongé de Pâques, les déplacements interrégionaux seront restreints à quelques motifs impérieux- ces motifs incluront évidemment les déplacements professionnels, mais aussi ceux liés à un motif familial, comme accompagner ou aller chercher un enfant chez un parent, un grand-parent ou un proche. Nous sommes en effet un gouvernement pragmatique et une certaine souplesse est toujours nécessaire pour permettre aux règles d'être mieux appropriées. J'observe du reste que l'immense majorité de nos concitoyens respecte spontanément les règles en vigueur, faisant preuve en cela d'un sens des responsabilités et d'un civisme qui les honorent. Mais je constate aussi avec vous qu'une minorité d'entre eux s'y refuse et je veux condamner devant vous sans réserve l'inconscience et l'irresponsabilité de certains qui se croient sans doute invincibles ou peut-être même immortels, alors que les ravages de la maladie nous démontrent chaque jour que personne n'est à l'abri du virus. Ces gestes inconséquents, qu'il s'agisse des rassemblements festifs, du non-respect du couvre-feu ou du refus du port du masque, doivent être prévenus et sanctionnés. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de l'intérieur d'accroître le nombre de policiers et de gendarmes affectés à cette tâche. Au lieu de s'occuper des voyous ! Nous veillerons notamment à ce que l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique soit strictement respectée. La consommation d'alcool dans l'espace public sera interdite. Très bien ! Sur arrêté préfectoral et en lien étroit avec les maires, l'accès à certains sites propices à des rassemblements en extérieur, comme des quais, des berges ou des places, pourra être interdit en fonction des circonstances locales. Il sera enfin demandé aux parquets de continuer à poursuivre systématiquement les auteurs de récidives portant sur l'organisation d'événements clandestins susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui. Pour autant, ces comportements ne doivent pas masquer, je l'ai dit et je le répète, la résilience et la haute conscience citoyenne de l'immense majorité des Français, partout sur le territoire, qui sans doute protestent, s'agacent des mesures et des freins mis à leur quotidien et s'interrogent, parfois à raison, mais qui se montrent respectueux des règles, c'est-à-dire finalement respectueux des autres. Autre décision forte que la situation nous contraint de prendre : fermer les établissements scolaires et les crèches et arrêter les activités périscolaires et extrascolaires. Tout a été fait, mesdames, messieurs les sénateurs, pour repousser au maximum cette décision. Je sais qu'il existait dans notre pays, comme dans cette assemblée, un très large consensus en faveur du maintien de l'accueil de tous les enfants dans les établissements scolaires. La France est du reste, vous le savez, le pays d'Europe qui a le moins fermé ses écoles. Rappelons en effet que les écoles sont restées fermées moins de 10 semaines en France depuis le début de la de la pandémie contre 24 en Allemagne, 26 au Royaume-Uni et 32 en Italie. Je crois que nous pouvons être fiers d'avoir maintenu cette exigence républicaine. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours considéré que, si nous devions- je ne m'en suis jamais caché devant vous -utiliser ce levier, il nous faudrait le faire en ultime recours et dans des conditions qui en réduisent le plus possible l'impact. Nous y sommes ! Les écoles, les collèges et les lycées ne sont pas épargnés par l'épidémie, et notamment par ce variant anglais. Depuis deux semaines, le taux d'incidence augmente plus vite chez les enfants et les adolescents que dans la population générale, ce qui a pour conséquence, dans le strict respect de nos propres normes sanitaires, de provoquer des fermetures de classes et d'écoles de plus en plus nombreuses. Nous devions donc reprendre l'initiative, en décidant que les établissements scolaires seront fermés pendant trois semaines, en optimisant, comme beaucoup l'avaient suggéré, la période des vacances de printemps, de sorte que les conséquences sur les enfants soient les moins pénalisantes possible. Concrètement, la semaine prochaine, où il n'y aura que quatre jours d'école, en raison du lundi de Pâques, tous les établissements scolaires assureront leurs enseignements à distance. Au cours des deux semaines suivantes, du 12 avril au 25 avril, tous les élèves de toutes les zones académiques seront en vacances dites de printemps, ce qui implique une modification du calendrier des vacances scolaires. Je mesure tout à fait l'impact de ces décisions sur la vie de nombreuses familles, mais aussi dans l'organisation des entreprises. Cependant, c'est le moyen d'atteindre notre objectif

Comme lors du premier confinement, un dispositif d'accueil des enfants des personnels prioritaires sera organisé dès la semaine prochaine, en lien avec l'éducation nationale et les collectivités locales. Les salariés qui seront conduits à garder leur enfant à domicile, faute d'autre solution, bénéficieront du dispositif d'activité partielle qui s'appliquait déjà lors du premier confinement. Il leur suffira de se signaler auprès de leur employeur, qui mettra en oeuvre la procédure de déclaration auprès des services compétents de l'État. Pour les élèves de l'enseignement supérieur, les règles en vigueur, qui prévoient un enseignement essentiellement en distanciel, seront maintenues, sans remettre en cause la possibilité donnée récemment aux étudiants de revenir une journée par semaine en présentiel, dans des conditions strictes. Je consulterai demain l'ensemble des associations d'élus locaux afin d'évoquer avec elles les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'ensemble de ces mesures, s'agissant notamment de la continuité des services publics et, en particulier, de l'accueil des enfants des personnels prioritaires. Bien évidemment, les dispositifs de soutien et d'accompagnement économique et social, dont le Sénat a bien voulu reconnaître l'intensité, tout en préconisant des améliorations, seront prolongés autant de temps que nécessaire. D'ores et déjà, certaines mesures ont été complétées, notamment en faveur des commerces fermés depuis février dans les grands centres commerciaux ou de ceux qui ont accumulé des stocks importants du fait des périodes de fermeture. Je pense également aux entreprises de plus grande taille affectées par de longs mois de crise. C'est le sens de l'aide exceptionnelle pour la prise en charge des coûts fixes, qui a été mise en place depuis hier, 31 mars. Les mesures que je vous présente cet après-midi sont difficiles, mais elles sont indispensables. Surtout, elles sont éclairées par la perspective de la campagne de vaccination, qui progresse et s'amplifie tous les jours, jours, nous donnant une vraie raison de penser que nous avançons sur la voie d'une sortie de crise. Plus de 8 millions de nos concitoyens sont désormais vaccinés, dont près de 2,8 millions avec deux doses. L'objectif de mon gouvernement reste le même : 10 millions de vaccinés à la mi-avril, 20 millions à la mi-mai et 30 millions à la mi-juin, en veillant bien sûr à ce que la Commission européenne fasse respecter les obligations des industriels quant au calendrier de livraison des doses. L'espoir fait vivre ! Nous serons donc au rendez-vous des objectifs que j'avais énoncés devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, le 17 décembre dernier, lors du débat organisé dans ce même hémicycle sur la stratégie vaccinale : j'avais alors annoncé la vaccination de 15 millions de personnes d'ici à la fin du premier semestre. Nous y serons très largement.

Surtout, nous sommes clairement les mieux positionnés pour la vaccination des personnes les plus vulnérables face à la maladie. Eh oui ! Je veux saluer toutes les personnes impliquées dans les centres de vaccination mis en place par les mairies, les établissements hospitaliers ou encore des professionnels de ville. Nous en comptons plus de 1 700 aujourd'hui, et d'autres encore doivent ouvrir dans les prochaines semaines. Je salue également la mobilisation des professionnels de ville : plus de 50 000 médecins et 20 000 officines de pharmacie se sont engagés dans la vaccination. En un mois, ils ont administré près de 1,7 million de doses aux patients éligibles. À compter de la semaine prochaine, 25 000 premiers infirmiers vont se lancer, à leur tour, dans la vaccination. Toujours la semaine prochaine, près de 1,4 million de doses supplémentaires seront utilisables sur le terrain, suivies de 3 millions de doses supplémentaires en avril et 3,6 millions en mai. Par ailleurs, vous le savez, le mois d'avril verra l'arrivée d'un nouveau vaccin, celui de Johnson & Johnson, qui a la particularité de ne nécessiter qu'une seule dose. Et Sanofi ? Il sera alors possible, dans les prochaines semaines, comme le chef de l'État l'a annoncé hier, d'ouvrir la vaccination à de nouvelles tranches d'âge : le 15 avril pour pour les personnes âgées de 60 ans à 69 ans ; le 15 mai pour les personnes âgées de 50 ans à 59 ans ; le 15 juin pour tous les autres. Nous travaillons également, en lien avec tous les secteurs professionnels concernés, à la réouverture prochaine des lieux et activités aujourd'hui fermés. Cette réouverture interviendra lorsque les conditions sanitaires seront réunies. Le moment venu, le Gouvernement présentera cette stratégie devant le Parlement. Il nous faut aussi nous prononcer, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les conditions d'organisation des élections régionales et départementales, prévues les 13 juin et 20 juin prochain. Ces élections ont déjà été reportées une première fois en raison de la covid-19. Encore un pari perdu ! Comme je l'ai déjà indiqué, et comme je le redis cet après-midi devant la Haute Assemblée, seules des raisons sanitaires impérieuses, de nature à compromettre l'organisation de la campagne ou du scrutin, pourraient justifier un nouveau report. En application de la loi du 22 février 2021, le conseil scientifique a rendu sur ce sujet un avis lundi J'observe avec vous que cet avis, particulièrement balancé, ne préconise pas explicitement un report des élections. C'est donc clairement le scénario de leur maintien que nous privilégions à ce stade. J'ajoute que les décisions dont nous débattons cet après-midi, y compris celles relatives à l'accélération de la vaccination, devraient avoir pour effet d'améliorer la situation sanitaire à l'échéance du mois de juin. ! ... le conseil scientifique formule des recommandations précises quant aux conditions de l'organisation et de la tenue de ces élections, tandis que les mesures nouvelles qui entreront en vigueur ce week-end, et pour quatre semaines, pourraient avoir un effet sur le déroulement de la campagne. Nous avons donc le devoir de de nous assurer que l'ensemble des conditions édictées par le conseil scientifique pourront être effectivement satisfaites et que leur mise en oeuvre très concrète ne viendra pas altérer l'expression libre et sécurisée du vote de nos concitoyens. À cet effet, je vais engager sans délai une consultation des partis politiques représentés au Parlement, parce qu'ils concourent à l'expression du suffrage, et des associations d'élus locaux, notamment les maires, chargés de l'organisation matérielle des opérations de vote. Un débat fondé sur l'article 50-1 de la Constitution sera ensuite organisé au Parlement, sur l'ensemble de ces éléments. Tel est le sens, monsieur le président

des semaines particulièrement difficiles sont encore devant nous. Plus que jamais, les personnels soignants, dont le dévouement et la bravoure sont admirables depuis quatorze mois, méritent notre soutien et la reconnaissance de la Nation tout entière. Je me rends très régulièrement dans les établissements de santé pour leur manifester ce soutien. Je sais, car ils me le disent, ce qu'ils endurent. Je sais combien ils se battent, malgré la fatigue, malgré la lassitude, pour sauver des vies. Notre système hospitalier va tenir le choc, et il va le tenir grâce à eux. Nous les y aiderons en continuant de mobiliser tous les leviers possibles : en déplafonnant les heures supplémentaires dans les établissements de santé en mobilisant tous les renforts possibles, en particulier les professionnels de ville, les retraités, les étudiants en santé, les 26 000 professionnels inscrits à la réserve sanitaire civile, mais également la réserve militaire en organisant la collaboration entre le public et le privé, qui n'a jamais été aussi fluide, j'y insiste ; en organisant des évacuations sanitaires depuis les régions les plus touchées. L'activation de l'ensemble de ces leviers doit nous permettre d'armer jusqu'à 10 200 lits de réanimation et d'accueillir tous les malades qui en auront besoin. Face à cette crise sans précédent et à la part d'incertitude que comporte cette épidémie,

Il y a évidemment, d'abord et en premier lieu, les critères épidémiologiques et sanitaires, et donc les avis des scientifiques et des médecins. Il me faut le dire et le répéter ici devant le Sénat et la Nation tout entière : il n'y a pas d'opposition entre le pouvoir politique et le pouvoir médical. Nous tenons le plus grand compte des avis, des analyses, des modèles et des prévisions des experts, conseils scientifiques et médicaux. Mais, et c'est bien là le rôle du Gouvernement, nous avons également le devoir- je dis bien : le devoir -d'intégrer dans nos prises de décision d'autres considérations, qui relèvent de la dimension sociale, scolaire, psychologique, économique de notre pays et de notre société. Ces critères se modélisent sûrement moins bien et leur impact est sûrement moins immédiat, mais leurs effets sont, un an après le début de la pandémie, beaucoup mieux connus. C'est dans la combinaison difficile, très difficile, de l'ensemble de ces critères que doit être recherché l'équilibre des décisions qu'il nous appartient de prendre. C'est aussi cet équilibre qui conditionne la temporalité de ces décisions. en fin de compte, et le moment dans lequel nous nous trouvons l'illustre parfaitement, la mère des priorités, le premier des critères qui finira toujours par s'imposer, c'est la protection sanitaire de nos concitoyens. Comme toujours, c'est dans l'unité et le recours aux valeurs de solidarité et de responsabilité que nous trouverons les ressources pour faire face à ce choc grave, inédit et complexe. C'est la caractéristique profonde de cette crise elle fait appel au sens des responsabilités de tous et de chacun. C'est cette responsabilité que je viens partager avec vous cet après-midi. Nous en

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Parlement est de nouveau saisi au titre de l'article 50-1 de la Constitution pour débattre des nouvelles mesures sanitaires annoncées hier soir par M. le Président de la République.

qu'il ne fallait pas revenir à un confinement dur, du type de celui que nous avons connu en mars 2020. Il nous paraît évident qu'un tel confinement ne serait plus accepté de la même manière par nos concitoyens. La peur et la sidération ont laissé place à l'inquiétude, la lassitude, et même parfois à une certaine colère. Cependant, l'évolution des indicateurs sanitaires imposait de nouvelles mesures.

Pour autant, ces mesures suscitent des interrogations que nous souhaiterions voir levées. D'abord, le passage d'une capacité de 7 000 lits à 10 000 lits en réanimation nous a valablement surpris. Alors que nous en parlons depuis des mois, comment cela est-il devenu réalisable ? On parlait d'« argent magique » ; aujourd'hui, nous avons des « lits magiques ». D'où sortent ces lits et pourquoi n'a-t-il pas été possible de les mobiliser avant ? Encore plus problématique est la question du personnel qui permettra de les faire fonctionner. Le Président de la République a bien précisé que tout le potentiel de la réserve sanitaire serait mobilisé, mais cela permettra-t-il de rendre effective l'utilisation de ces nouveaux lits ? J'en viens à la stratégie vaccinale. Jusqu'ici, outre les seniors, seuls les soignants étaient prioritaires pour se faire vacciner. À notre sens, l'ouverture de cette priorité à de nouvelles catégories, à savoir les enseignants, les policiers ou les pompiers,

De même, pourquoi pas les chauffeurs de bus ou les caissières de supermarché, dont on a tant parlé voilà quelques mois ? N'y a-t-il pas là un risque de revendications tous azimuts et d'incompréhension de la part d'un certain nombre de professions exposées ? Toujours au sujet des vaccins, mais cette fois en amont, au niveau de la production et de la fourniture des doses, les annonces présidentielles sont très volontaristes et optimistes. Vous avez dit que nous allions accélérer les achats. On ne peut qu'être d'accord, mais tout un chacun sait bien que les doses manquent.

Le chef de l'État n'a pas parlé des autotests, alors qu'ils sont très utilisés en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pourquoi faisons-nous l'impasse en France ? Pourquoi avons-nous été moins réactifs que nos voisins européens pour nous en équiper ? Autre grand absent du discours présidentiel, le pass sanitaire. C'est pourtant un sujet majeur, aux niveaux tant communautaire que national. Toutes les restrictions sanitaires seront-elles levées une fois que les publics à risque auront été vaccinés ? Enfin, on peut se demander s'il n'aurait pas été possible de conserver au moins un peu de différenciation locale, s'il n'aurait pas été envisageable de jouer la carte de la déconcentration et de plus inciter les praticiens hospitaliers à innover. Vous l'aurez compris, monsieur le Premier ministre, il s'agit là d'interrogations. Elles ne remettent pas en cause l'idée que nous nous faisons de votre action. Il ne s'agit pas d'exprimer une forme de défiance ni de mettre en doute la bonne foi du Gouvernement, pas plus que de contester l'idée que vous défendez la protection sanitaire des Français tout en ménageant autant que possible les autres intérêts de la Nation. Vous avez parlé des aides économiques. Chacun ici peut constater que le Gouvernement, l'État, a fait beaucoup ces derniers mois pour aider les entreprises, les commerçants. Cependant, nous ne voterons pas cet après-midi, monsieur le Premier ministre, car, une fois de plus, nous débattons de mesures déjà prises.

révèle un problème institutionnel, monsieur le Premier ministre. C'est de cela que nous voulons vous parler aujourd'hui. Les mesures sanitaires vont dans le bon sens, mais on prend des mesures qui touchent aux libertés publiques. Vous avez dit ce matin que votre action se faisait naturellement dans un cadre constitutionnel, mais surtout à travers des mesures administratives

Il n'y a rien d'offensant, monsieur le Premier ministre, ni pour le Président de la République ni pour votre gouvernement, à ce que les parlementaires puissent émettre une opinion ou formuler des recommandations.

aujourd'hui ? S'il est devenu un corps central, indispensable dans l'action qui est menée aujourd'hui, le Parlement, lui, a disparu de la prise de décision. On va même jusqu'à créer des « machins machins »- le général de Gaulle les aurait appelés ainsi -, avec un certain nombre de citoyens tirés au sort pour savoir ce qu'ils pensent des difficultés vaccinales. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne les entend plus ... Le Président de la République a décidé de parler directement à l'opinion. Je pense que c'est un exercice très dangereux, comme on a pu en faire l'expérience avec l'épisode des « gilets jaunes ». Cela paraît déjà très loin, mais c'est finalement très récent.

Vous aviez précédemment déclaré que vous vous appuieriez sur les conclusions du conseil scientifique. Je reconnais, comme vous, que celles-ci sont « balancées

! » Évidemment, monsieur le Premier ministre, il va falloir trouver d'autres éléments. Pour notre part, nous considérons qu'il y a des dates électorales, des modes de scrutin, et que, sauf événement extrêmement extrêmement important, il n'y a pas lieu de modifier le processus. Mon dernier point, monsieur le Premier ministre, porte sur l'Europe. Beaucoup des sujets dont nous parlons relèvent de l'action européenne. avons déjà eu l'occasion d'en parler ici, notamment au moment des questions d'actualité au Gouvernement. Le plan de relance nous inquiète, parce qu'il y aura aussi

le 29 octobre dernier, vous veniez déjà devant nous pour annoncer des mesures nécessaires au vu de l'évolution de la situation sanitaire. J'avais souligné la difficulté de votre tâche, ainsi que la responsabilité qui était la vôtre devant les Français. Malgré les errements, malgré les fautes, malgré la trop grande verticalité de votre gestion de crise, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avait voté en faveur de votre déclaration. Notre vote ne valait pas soutien à l'action de votre gouvernement. Notre vote ne valait pas quitus pour votre gestion de la crise. Nous avions voté en faveur des Français et de leur santé. Cinq mois plus tard, la situation a changé, ou, plutôt, elle n'a pas changé. Vous n'avez pas tiré les enseignements des précédentes séquences. La gestion de l'épidémie s'est dégradée. La concentration du pouvoir s'est renforcée. Cinq mois plus tard, vous êtes devant nous et nous ne savons pas pourquoi, monsieur le Premier ministre. En déclinant les propos de l'oracle présidentiel, vous ne nous associez pas. Le vote du Parlement serait unanimement défavorable que cela ne changerait rien Cela fait des mois que nous vous demandons plus de transparence, plus de clarté, plus de démocratie sanitaire. Cela fait des mois que vous balayez d'un revers de main nos nombreuses propositions. Cela fait des mois que vous prenez les chambres parlementaires pour un paillasson au service de la doxa élyséenne. Le Parlement vote ... Oui, il vote, quand il a discuté un texte, un texte qu'il a travaillé, un texte qu'il a amendé. Là, on ne discute de rien ; on n'amende rien. On acclame ou on conspue. C'est toujours le même schéma : le bunker du conseil de défense suffit ; la parole du président suffit ; le Premier ministre répète et le Parlement enregistre. Vous me pardonnerez donc, monsieur le Premier ministre, que mon intervention se fonde sur l'intervention du Président de la République plutôt que sur la vôtre. Le Président de la République, hier soir, a tenu à justifier son action pour éviter tout. Si certaines erreurs ont été confessées du bout des lèvres, aucun mot n'a été prononcé pour les morts de la pandémie, ou si peu. Pour combler ce manque, je tiens à avoir une pensée pour nos compatriotes qui ont été touchés par ce virus, avec parfois des conséquences sur le long terme, pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui se battent actuellement contre cette maladie. Bientôt, plus de 100 000 des nôtres ne seront plus à nos côtés- probablement davantage, si l'on compte les effets des nombreuses déprogrammations dans nos hôpitaux. Nous payons aujourd'hui les conséquences des choix du Président de la République. Il faut le dire ! Il décide seul, il doit assumer seul. Il dit avoir gagné du temps de liberté pour les Français, mais de quelle liberté parlons-nous ? Depuis la fin de janvier, chaque semaine, les Français sont en alerte devant les rumeurs d'une intervention présidentielle. Chaque semaine ou presque, de nouveaux territoires sont touchés par des restrictions. L'exécutif s'est félicité pendant de longs mois, déraisonnablement, de ne pas avoir écouté les scientifiques, qui préconisaient des mesures de freinage plus fortes dès la fin de janvier en raison de l'apparition des variants. Pourtant, la flambée annoncée a bien eu lieu : nous sommes en plein dedans Ainsi, sans y associer le Parlement ou les Français, votre gouvernement applique la décision du Président de la République en laissant le virus circuler à un niveau élevé depuis deux mois. Pourtant, le conseil scientifique avait indiqué à la fin de janvier : « Si nous ne réussissons pas à endiguer la progression du virus avec des mesures fortes, nous risquons d'être confrontés à des pics épidémiques similaires à ceux observés en mars-avril et novembre 2020, voire plus élevés. » Vous-même, monsieur le Premier ministre, le 28 janvier, lors d'un fameux comité de liaison parlementaire, alors que le variant anglais ne représentait que 10 % des infections, vous nous affichiez des projections qui montraient un emballement inévitable de l'épidémie. Ces

l'épidémiologiste en chef, celui pour qui aucun sujet n'est inaccessible au vu de son intelligence hors du commun, en a décidé autrement ! Le pari du « trou de souris » du Président de la République est perdu. Qu'il le dise, qu'il l'assume, qu'il s'excuse, car cela aurait pu être évité ! Lui qui voulait écarter la perspective d'une dictature sanitaire a provoqué une débâcle. Le résultat de cette débâcle est un nouveau confinement et le tri des patients. Voilà deux termes que l'on n'entend pas, encore aujourd'hui, dans la bouche des membres de l'exécutif : « confinement » et « tri ». Mais ce n'est pas parce que l'on ne nomme pas les choses qu'elles n'existent pas. Quand on restreint la liberté de circulation, quand on ferme les écoles, quand on ferme les commerces, on confine Quand on déprogramme massivement des opérations, on trie ! Non ! Cette politique résulte du choix fait par un homme, dans une démarche de concentration excessive de ses prérogatives constitutionnelles. Je le rappelle à cette tribune : la politique de santé ne fait pas partie du domaine réservé du Président de la République

Nous connaissons la complexité d'une telle crise, nous ne nions pas les difficultés de gestion qu'elle entraîne et nous sommes toujours prêts à agir à vos côtés, mais il faut nous en donner la possibilité. Dès cet automne, nous vous avons interrogé sur l'organisation de la stratégie vaccinale, notre seul espoir pour sortir de cette crise sanitaire. Nous appelions le Gouvernement à mettre en place rapidement un plan clair, net et précis de vaccination. Ce n'était pas de la polémique, mais un appel à la prise en compte de l'urgence absolue par l'exécutif. Vous étiez rassurant, vous nous affirmiez que vous étiez dans l'action, alors que quelques semaines plus tard vous n'avez été que dans la réaction ! C'est le dos au mur que vous réagissez, comme d'habitude, comme aujourd'hui. Ce retard a un coût économique, social et humain important. Ce manque d'anticipation, associé à une stratégie assumée de la lenteur, à laquelle vous avez heureusement renoncé, doit s'effacer au profit d'une mobilisation générale que vous annoncez, mais qui ne se traduit pas encore dans les chiffres. Voici le résultat : en France, seule 13 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Nous sommes au-delà de la vingtième place des pays qui vaccinent le plus. Je connais votre argument, monsieur le Premier ministre : notre situation n'est pas pire qu'ailleurs. Non, elle est meilleure ! Votre position me fait penser à cet adage québécois bien connu : « Quand on se regarde, on se désole ; quand on se compare, on se console. » Monsieur le Premier ministre, nous ne voulons pas être consolés ; nous voulons être les plus performants et tout faire pour que l'Europe ne soit pas le bouc émissaire de ces difficultés. Le 3 décembre dernier, vous nous annonciez que 15 millions de personnes seraient vaccinées avant le printemps, soit la fin du mois de mars. Non ! Nous y sommes : 8 millions de personnes ont reçu une dose, soit la moitié de ce que vous aviez annoncé. Les retards de livraison n'expliquent pas tout. de la désorganisation ? des volte-face sur les vaccinodromes ? Hier soir, le Président de la République a annoncé de nouvelles arrivées de vaccins, ainsi que la production de vaccins en France. Tant mieux, mais donnez-nous des chiffres, montrez-les-nous, expliquez-nous comment vous allez réaliser cela. C'est ainsi qu'on associe à son travail le Parlement et les Français. Hier soir, le Président de la République a annoncé un plan de sortie de crise. Il aurait pu parler de déconfinement, comme au printemps dernier. Sur ce sujet, je ferai les mêmes requêtes : donnez-nous des chiffres, montrez-les-nous, expliquez-nous Comment vous croire, alors que le Président de la République ou le porte-parole du Gouvernement, dans un savant mélange de Madame Irma et de Pinocchio, annonçaient un retour à la vie normale à la mi-avril et que nous discutons aujourd'hui d'un confinement auquel vous êtes maintenant acculé, pour ne pas avoir su l'anticiper ? Hier soir, le Président de la République a annoncé de nouveaux lits de réanimation. Comment monter à 10 000, alors qu'il y a moins d'un an vous en promettiez beaucoup plus et que vous n'avez pas pu tenir vos promesses ? Comment vous faire confiance aujourd'hui quand les soignants sont à bout et que le Ségur de la santé a changé si peu de choses ? Ce n'est pas vrai ! Les mesures que vous prenez aujourd'hui sont nécessaires, nous regrettons qu'elles arrivent trop tard et que votre procrastination sanitaire empêche de continuer une politique territorialisée que vous avez mis bien du temps à mettre en place, malgré les demandes des élus locaux. Avoir laissé les écoles ouvertes est effectivement une fierté pour notre pays. Nous regrettons qu'il faille les fermer aujourd'hui, sans que les tests salivaires aient été livrés ou que la continuité pédagogique ait pu être facilitée par des investissements qui auraient permis de surmonter la précarité numérique de nombreux élèves.

Par ailleurs, le ruissellement de la dette publique sert d'amortisseur économique et social. Nous avons soutenu vos décisions, mais nous voulons savoir comment aller plus loin, alors que la crise révèle et exacerbe les inégalités, mais que vous n'entendez pas nos propositions statut des travailleurs précaires, fracture numérique et éducative, aide alimentaire, situation des étudiants les plus fragiles. Nous avons demandé que l'on prévienne le risque d'accroissement des situations de précarité et de pauvreté. Le RSA pour les moins de 25 ans : rejeté ; le débat sur le statut des travailleurs des plateformes : rejeté ! Pour éviter d'accroître encore la précarité et les inégalités, nous avons proposé des solidarités fiscales nouvelles, des fonds des fonds de soutien, des orientations ciblées pour le plan de relance en faveur des ménages les plus fragilisés. Quand nous proposons une réévaluation des aides au logement et la suppression de la réforme de ces mêmes aides, qui pénalise les jeunes qui entrent sur le marché du travail, vous répondez par la relance de la réforme de l'assurance chômage. Nous avons fait des propositions visant à préserver l'activité locale de proximité, en demandant un traitement différencié et une meilleure concertation avec les élus locaux pour pallier le manque de confiance des commerçants dans les aides de l'État ; rien n'a changé ! L'économie de proximité doit être mieux identifiée comme une priorité de la relance ; rien n'a été retenu par votre gouvernement. Pour ne pas confiner la démocratie, monsieur le Premier ministre- vous avez évoqué ce sujet à la fin de votre discours -, nous avons également proposé, à de multiples reprises, des mesures qui permettent la tenue des scrutins départementaux et régionaux dans les meilleures conditions, mesures d'ailleurs recommandées dans le rapport du conseil scientifique.

Vous avez voulu freiner pour ne pas enfermer, mais vous devez maintenant enfermer pour freiner, alors que le train de la covid-19 est lancé à pleine vitesse : 40 000 à 50 000 cas par jour Votre gestion de la crise est un jour sans fin pour la France. Les Français ne sont pas résilients, monsieur le Premier ministre : aujourd'hui, ils sont résignés. Ils attendent autre chose. L'annonce de la lumière au bout du tunnel, tellement invoquée, nous amène à nous interroger sur la crédibilité de votre stratégie et, peut-être plus encore, sur celle de votre stratège. Vous avez accepté que nous vivions avec le virus, alors que nous aurions dû nous donner comme objectif de l'éradiquer au plus vite. Face à cette parodie politique, face à cette mascarade de démocratie, face à ce simulacre de concertation, nous avons décidé de ne pas être les faire-valoir de l'exécutif. Le Sénat ne disposant pas du pouvoir de censure,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, hier soir, le président Macron a confessé ce que les Français savaient déjà depuis longtemps, pour en avoir subi les conséquences graves : il a confessé qu'il avait « commis des erreurs erreurs ». Voyez-vous, monsieur le Premier ministre, le problème est que vous en commettez encore et que leurs conséquences ne seront pas moins importantes que celles des précédentes, notamment en matière de promesses non tenues sur la création de lits en réanimation. Nous avons également entendu dire hier soir que « l'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas miner les efforts de tous ». Les Français seraient-ils encore montrés du doigt, ou le Président parlait-il tout simplement de votre gouvernement ? Face à l'offensive du variant anglais, toutes ces nouvelles mesures liberticides sont les conséquences directes du Waterloo de la vaccination, qui marque la déroute de votre gouvernement.

Vous, vous êtes en retrait, en retard, et chaque jour la bataille de la vie est perdue pour des dizaines, voire des centaines de nos compatriotes. Vous n'avez qu'un horizon à offrir à notre peuple : promettre des lendemains qui enferment ! Vos annonces condamnent les étudiants et les plus jeunes à la détresse, les ouvriers à rester exposés, les indépendants et les commerces de proximité, dont il est scientifiquement reconnu qu'ils ne constituent nullement un lieu de contamination, à fermer définitivement. Quant à la mère ou au père qui va pouvoir télétravailler, il devra « en même temps faire la classe à son enfant, voire à ses enfants. On lui souhaite beaucoup de courage et d'abnégation ! La dette est si abyssale qu'elle va se transformer en trou noir, car votre confinement coûte à la France, selon Bercy, 365 millions d'euros par jour Nos compatriotes sont condamnés à être tributaires d'un calendrier de la vaccination très incertain en raison, entre autres choses, de votre « poutinophobie », qui vous pousse encore à refuser le vaccin russe que les Allemands et les Italiens ne se privent pas de commander par millions. Et que dire de l'absence totale, voire du rejet de tout traitement qui permettrait de contenir la flambée d'hospitalisations ! Je pense au traitement du professeur Raoult, à Marseille, traitement qui avait pour seul tort non pas d'être dangereux, mais de soigner quasiment gratuitement un véritable cauchemar, un virus, un empêcheur de se goinfrer en rond pour les grands laboratoires ! Le professeur Raoult a été banni en même temps que son traitement, dont nombre d'élus marseillais et personnalités de haut rang ont pu bénéficier

de la liberté de décision. En ces temps d'enfermement tous azimuts, la vérité nous rend libres. Or, à la vérité, le retour- la résurrection, si j'ose dire -de nos libertés n'est annoncé ni pour dimanche, ni pour lundi, ni pour les semaines à venir. je ne saurais cautionner cet enfer économique, social et autoritaire dans lequel vous souhaitez enfermer le pays un mois de plus.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, une fois de plus, la vague est montée ; une fois de plus, l'hôpital est submergé ; une fois de plus, le Président a parlé ; une fois de plus, le Parlement est pris en otage ; une fois de plus- la troisième -, la France est confinée. Monsieur le Premier ministre, dans quelques instants, vous allez nous demander de voter, mais ce sera un vote pour rien, parce que c'est un vote sur rien. Vous allez nous demander de voter sur des annonces qui ont déjà été faites ; vous allez nous demander de voter sur des mesures à prendre qui ont déjà été prises

La contrepartie de ces pouvoirs immenses serait de veiller au contrôle démocratique et notamment parlementaire. Pour autant, vous vous ingéniez méticuleusement à marginaliser le Parlement.

La démocratie consiste à rendre des comptes. Aux heures les plus graves de notre histoire, pendant la Première Guerre mondiale- relisez votre histoire ! -, cette démocratie n'a pas été un obstacle à la gestion d'une crise énorme : elle a été une ressource. Or quels sont ces mécanismes qui se mettent en place ? Ce sont les réseaux sociaux, où chacun

le Premier ministre, qui êtes chargé de la protection des Français, de la nation française ; aucun commissaire européen ne fera pour le peuple français ce qu'un élu du peuple

Ce geste politique n'est pas un mouvement de mauvaise humeur ou un caprice, mais tout simplement un message : la démocratie représentative, c'est l'assurance pour tous les Français, quels qu'ils soient

monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis l'annonce inespérée de la découverte de vaccins en quelques mois seulement par des chercheurs que nous ne remercierons jamais assez, la course est lancée entre l'acquisition de l'immunité collective qui nous sauvera de la pandémie et la dissémination des nouveaux variants du virus qui signerait notre défaite. Cette équation à deux inconnues est une ordalie pour le Gouvernement comme pour les Français, parce qu'elle se complique de deux paramètres qui en font l'effroyable complexité. Le premier est le retentissement immédiat de toute mesure sanitaire sur l'économie du pays qui, dans le cas extrême d'un confinement total, s'écroule aussitôt, nous l'avons vécu. Le second est le désastre psychique causé par une crise interminable pour tous nos concitoyens, dont beaucoup sont désormais au bord de l'effondrement, ou tout au moins de l'épuisement. Jamais la situation n'a été aussi tendue ; c'est pourquoi, même si nous entrevoyons la lumière au bout du tunnel, nous sentons tous que les semaines qui viennent seront cruciales. C'est sans doute la raison pour laquelle la décision du Président de la République de ne pas reconfiner en janvier dernier, mais de prendre des mesures graduelles, s'exemptant pour la première fois des injonctions scientifiques, a été très majoritairement approuvée par les Français, malgré ceux qui ont souligné les risques, les insuffisances ou l'aspect hasardeux de ce pari. Je le dis clairement : je fais partie, avec beaucoup d'autres ici, de ceux qui ont approuvé cette stratégie et je ne peux donc aujourd'hui critiquer le Président de la République en me demandant s'il n'aurait pas dû prendre il y a deux mois les décisions qu'il prend ce jour, voire des décisions plus radicales encore. Ce serait oublier aussi que, depuis des mois, les enfants sont allés à l'école, que les entreprises ont tourné et que la plupart des Français on put mener une vie presque normale serait oublier encore que, en raison des nouveaux variants, la certitude d'une efficacité absolue d'un confinement n'était pas acquise, contrairement à l'année dernière. Avec des mesures plus radicales que les nôtres depuis deux mois, l'Allemagne est aujourd'hui quasiment au même nombre de décès quotidiens que nous, l'Italie en a presque le double. Très bien ! Le même dilemme se pose aujourd'hui avec une intensité décuplée par des courbes qui remontent, par des critiques qui fusent de nouveau et, enfin et peut-être surtout, par les pressions pour des mesures radicales d'une partie du corps médical, peut-être déçue que l'on ne suive plus ses prescriptions à la lettre. Loin de moi la prétention de nier les difficultés extrêmes, et qui s'aggraveront dans les jours qui viennent, que connaissent les services de soins intensifs, loin de moi l'idée de minimiser le dévouement inlassable des soignants, dont beaucoup sont, eux aussi, au bord de l'épuisement, mais il faut rendre à César ce qui est à César et au politique ses prérogatives. La première d'entre elles est la responsabilité de juger des moyens de tenir dans l'adversité, l'adversité, en prenant en compte les préoccupations, les possibilités, les capacités de résistance ou les cauchemars de tous les Français, en ayant à l'esprit que le choix est rarement entre une bonne et une mauvaise solution, entre une mauvaise solution et une autre, pire encore. Ce choix est d'autant plus difficile que les médecins eux-mêmes sont partagés, il suffit de regarder les plateaux de télévision, de jour comme de nuit, pour s'en convaincre.

un patron de la Pitié-Salpêtrière appelait avant-hier à la fermeture immédiate des écoles ; la Société française de pédiatrie lui répondait le lendemain qu'il fallait tout faire pour éviter de fermer des écoles. C'est dans ce contexte que le Président de la République a dû prendre une décision que j'imagine déchirante. Camper sur des mesures dont il apparaît désormais qu'elles ne suffisent plus à réduire l'épidémie, c'était la certitude de perdre la course de vitesse contre le virus ; reconfiner totalement, c'était une capitulation, prendre aussi le risque d'une révolte d'une partie de nos concitoyens, nous le voyons tous dans nos départements. L'exécutif a choisi l'accentuation des mesures de freinage plutôt que le retour à un confinement strict étendre à l'ensemble du territoire métropolitain les mesures qui prévalaient déjà dans les territoires les plus touchés et prolonger les vacances scolaires de quinze jours tout en laissant ouvertes les crèches et les écoles Ces mesures seront sans doute douloureusement ressenties dans des régions qui pouvaient se sentir à l'abri, mais qui, en réalité, et chaque jour nous le démontre un peu plus, ne le sont pas, par des commerçants déjà durement éprouvés et par des parents épuisés, se demandant comment ils pourront concilier profession et garde des enfants elles seront en réalité ressenties douloureusement partout, mais je ne vois guère d'alternative. La clé de notre avenir, ce sont désormais les vaccins et, surtout, la campagne pour les délivrer. Le début de cette campagne a donné lieu à beaucoup de critiques, sur sa lenteur, sur la décision de s'en remettre à l'Europe, sur la

j'ai dit à plusieurs reprises qu'il fallait aller plus vite, que le principe de précaution ruine parfois ceux qu'il prétend défendre et que ma crainte n'était pas que les vaccins restent dans les congélateurs, mais, au contraire, qu'il n'y en ait pas assez. République, dans son discours d'hier, a pris la mesure de cet enjeu crucial. L'accélération est impérative, nous devons nous donner les moyens d'y parvenir. Le Gouvernement n'a désormais d'autre choix que de réussir. Le succès de la vaccination est entre les mains de l'exécutif, tenu à une obligation de résultat. Il sait qu'il peut compter sur l'ensemble des élus locaux, qui ne cessent de faire la preuve de leur dévouement et de leur efficacité. Plusieurs groupes de notre assemblée ont annoncé leur intention de ne pas participer au vote qui conclura ce débat. Je comprends leur agacement et, pour certains, leur irritation. La V République n'est pas tendre pour le Parlement et ce n'est pas la première fois que nous nous plaignons de la façon dont nous sommes traités par l'exécutif. Toutefois, la question qui nous est posée aujourd'hui est d'une telle importance pour l'avenir de nos concitoyens, pour les mois et, peut-être, pour les années à venir, pour notre santé, pour notre économie, pour notre futur en un mot, qu'il ne nous paraît pas possible, en plein milieu de la pire crise sanitaire depuis des années, de ne pas prendre nos responsabilités. Les Français ont le droit de connaître l'opinion de leurs élus lorsque l'essentiel est en jeu. C'est la raison pour laquelle nous participerons à ce scrutin. C'est toujours lorsque l'on est sur le point de réussir que la tentation de renoncer est la plus forte c'est toujours le dernier effort qui est le plus douloureux ; c'est celui qui nous est demandé aujourd'hui. Pour la première fois, il est accompagné d'un message d'espoir crédible qui permet de fixer des échéances précises et annoncées. Cette crise est une épreuve, mais ce n'est qu'une épreuve et l'humanité en a surmonté de bien plus graves. Dans quelques mois, grâce aux vaccins, grâce à notre respect des règles, grâce à notre solidarité, 2021 sera l'année où nous surmonterons à notre tour l'épreuve qui nous est assignée. La parole

un an de pandémie et 4,6 millions de malades ; un an de pandémie et un personnel soignant à bout de souffle ; un an de pandémie et des inégalités sociales qui explosent un an de pandémie et plus de 10 millions de pauvres dans notre pays ; un an de pandémie et une entreprise sur trois menacée de faillite, malgré les aides gouvernementales ; un an de pandémie et de détresse psychologique ; un an de pandémie et une jeunesse aux abois un an de pandémie et une vie sociale et culturelle sous cloche ; un an de pandémie et des perspectives toujours aussi incertaines. Le bilan sanitaire, social et économique du covid-19 est dramatique et ses conséquences se feront ressentir pendant des années.

mais il n'est pas non plus possible de vous exonérer de votre responsabilité, et en particulier d'exonérer le Président de la République de la sienne. Monsieur le Premier ministre, je relisais les propos que j'ai tenus lors du débat organisé dans de pareilles circonstances le 29 octobre dernier et cette lecture m'a désespéré rien n'a changé depuis un an, rien n'a changé depuis cinq mois. Jupiter l'épidémiologiste, Jupiter le roi thaumaturge, Jupiter le maître des horloges décide de tout, tout seul, et vous venez ensuite faire le service après-vente devant nous.

Vous n'avez pas su construire l'union nationale, indispensable à la période. Rien n'a changé et le Président de la République continue vainement de l'invoquer comme on crie dans le vent. opportun et intelligent d'associer la représentation nationale aux décisions permettant de faire face à la situation sanitaire, économique et sociale, tout en protégeant les libertés individuelles. C'est comme cela que fonctionne une démocratie normale. Si l'on avait encore un doute quant au fait que la V République n'est pas une démocratie normale, celui-ci est levé depuis un an ! Le Parlement aurait dû retrouver toute sa place, il était dans votre intérêt, dans notre intérêt collectif, d'associer réellement l'opposition aux prises de décisions. Encore moins que d'habitude, l'exécutif ne peut avoir raison tout seul. La complexité du défi auquel nous faisons face aurait nécessité, et nécessite toujours de s'appuyer sur l'intelligence et sur la responsabilité collective des élus du peuple plutôt que sur l'intelligence d'un seul homme- aussi supérieure soit-elle -, qui n'est responsable devant personne, selon notre bancale Constitution. En la matière, vous auriez également dû associer beaucoup plus étroitement les élus locaux. Hélas, la consultation des territoires au préalable de décisions d'ampleur nationale comme celles que vous présentez aujourd'hui est toujours inexistante. Quand les élus sont responsables et de bonne composition à votre endroit, je pense par exemple au maire de Lyon, vos ministres les récompensent par des accusations fallacieuses et des polémiques médiocres, au lieu de consacrer leur temps et leur énergie à la résolution de la crise. La gouvernance demeure solitaire et erratique. Ce manque total de visibilité affaiblit chaque jour davantage l'acceptabilité des mesures qui sont prises et leur efficacité. C'est un cercle vicieux qui nous dessert toutes et tous collectivement. En un an, vous n'avez jamais été capables de donner de la visibilité aux Françaises et aux Français. Certes, la situation est instable et difficilement prévisible, mais d'autres pays ont fait beaucoup mieux, je pense notamment à l'Afrique du Sud, pourtant très durement touchée par le virus, qui a pris le temps d'élaborer un mode de gouvernance intéressant. En lien avec le parlement, le gouvernement y a mis en place un barème à cinq niveaux d'alerte, à la manière de notre barème Vigipirate. À chaque niveau correspond progressivement un certain nombre de mesures de distanciation et de restriction de la liberté de mouvement et d'activité. Le changement de niveau est activé par le gouvernement, sur la base de critères objectifs : circulation du virus, nombre de décès, niveau d'occupation des hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui empêche le Gouvernement de mettre en place un tel dispositif, qui permettrait de donner de la visibilité aux Françaises et aux Français, aux élus locaux et aux entreprises, de renforcer l'acceptabilité des mesures et de soulager notre démocratie ? Enfin, qu'est-ce qui empêche également de demander à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), comme l'ont d'ailleurs fait aussi l'Afrique du Sud et l'Inde, la levée des brevets sur les vaccins, car pour vacciner, il faut des vaccins et il faut en produire. Ce constat longuement posé, c'est désabusé et sans grand espoir que vous entendiez mon message que je vais néanmoins formuler quelques demandes pour accompagner les mesures que vous présentez cet après-midi et dont je ne conteste pas, faute d'alternative, le bien-fondé. Il faut, d'abord, renforcer les moyens de l'hôpital. Le Ségur de la santé est insuffisant, les soignants sont exsangues, on peine à recruter des infirmières et des infirmiers. Il faut les récompenser davantage pour les efforts de la période et revaloriser leurs salaires de manière pérenne et significative. Il faut aussi renforcer les moyens matériels et humains. Le Président de la République promettait jusqu'à 12 000 lits de réanimation en octobre, nous en sommes, selon ses dires, à 7 000. À Lyon, à Bordeaux, les hôpitaux militaires ferment alors qu'ils auraient pu accueillir des malades. Monsieur le ministre, entendez enfin la lassitude et l'exaspération des soignants sans lesquels le bilan de la pandémie serait catastrophique. Comment cette crise n'a-t-elle pas encore débouché sur un plan Marshall pour l'hôpital public ? D'autre part, il est plus que temps de prendre des mesures d'urgence sociale dignes de ce nom. Nous avons déjà des mois de retard : 10 millions de pauvres, des étudiants qui vont à la soupe populaire, votre dogmatisme néo-libéral est incompréhensible. Il faut abroger la réforme de l'assurance chômage, augmenter les minimas sociaux et automatiser leurs versements, élargir le RSA aux moins de 25 ans, rétablir les contrats aidés, aider les associations et tendre, demain, vers un revenu universel. Nous vous demandons également une vigilance accrue envers tous les publics exposés par le confinement : les personnes seules, les personnes psychologiquement fragiles, les victimes de violences conjugales, tout particulièrement les femmes. Vous fermez les écoles un mois, le temps des vacances de Pâques. Nous vous faisions cette proposition la semaine dernière, lors des questions au Gouvernement ... Exact ! Nous sommes aujourd'hui soulagés que l'évidence ait fini par s'imposer. Le retard de la vaccination explique, en partie, cette situation et les personnels scolaires doivent devenir un public prioritaire, car le manque de moyens, notamment humains, et les difficultés à trouver des remplaçants en sont aussi de la République évoquait le « combat du siècle » à propos du décrochage scolaire et des retards d'apprentissage de notre jeunesse. Espérons que, pour une fois, il ne s'agisse pas de ces propos incantatoires dont il a tant l'habitude,

Enfermé dans votre idéologie, vous vous y refusez depuis le printemps dernier, pourtant, c'est indispensable d'un point de vue financier comme d'un point de vue moral pour garantir l'unité du pays. Il faut mettre en place une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont la richesse s'accroît encore malgré la crise. Il en faut une autre sur toutes les entreprises qui ont fait des bénéfices grâce à la crise, notamment les géants de la vente en ligne et les grandes surfaces. Monsieur le Premier ministre, les écologistes n'ont cessé d'être constructifs durant cette crise qui nous engage toutes et tous. Nous continuerons à l'être, quand vous voudrez bien nous consulter en amont. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, je le regrette, et vous comprendrez que nous ne prenions pas part, non plus, à cette mascarade démocratique. La

au-delà des talents d'orateur qu'ont déployés ceux qui m'ont précédé, la dureté de certains propos, la véhémence de certaines attaques, les sarcasmes faciles, les procès sans appel

Cela fait un an que l'inquiétude du covid-19 frappe l'ensemble des pays du monde, bouleversant les échanges, endeuillant les familles, transformant nos vies. Chacun d'entre nous a vécu dans sa ville, dans son entourage, dans son intimité, le doute, l'éloignement, la solitude et parfois le décès. Un an pour mieux comprendre ce virus nouveau, c'est désormais le cas ; un an pour s'armer face à lui, pour lutter, chacun, mois par mois, contre l'évolution de la maladie, avec, en perspective, la vaccination en première ligne ; un an nous avons tous dû prendre, en conscience, des décisions cruciales avec pour objectif d'agir en responsabilité et, pour nous tous, de tenir ensemble. La question qui nous est posée aujourd'hui, après l'Assemblée nationale, est d'apporter ou non notre adhésion aux mesures prises par le chef de l'État et par le Gouvernement.

vous tombez dans une irresponsabilité qui vous déshonore quelque peu. Il y aura eu bien des anathèmes, bien des mises en demeure,

il existe une multitude de réalités, des parents débordés, des enfants seuls face à leurs difficultés, d'autres, entourés par des tuteurs. En laissant les écoles ouvertes, monsieur le ministre de l'éducation nationale, pendant 42 semaines, le choix a été fait de pallier ces inégalités, ce qui nous préserve aujourd'hui

Merci, mes chers collègues, ces applaudissements me font chaud au coeur ! Pourrions-nous enfin sortir du jeu politique et des postures binaires qui, trop souvent, dénaturent notre débat ? Notre rôle impose que chacun de nos mots soit choisi avec responsabilité, dans ce climat où il est si facile de les user comme des leçons, des reproches ou des menaces. J'entends qu'il y aurait d'un côté, ici ou là, ceux qui critiquent, qui savent, qui prédisent, qui écoutent et qui ne décident jamais et, de l'autre, ceux qui ignorent, qui sont arrogants, qui ne consultent pas, qui n'entendent pas, qui décident et dont les décisions sont toujours contestées. ce jeu-là ne fait pas avancer notre pays, non plus que la lutte contre le virus. Nous pouvons en sortir, parce que l'expérience de cette année de drame épidémiologique nous a apporté un certain nombre d'enseignements. Quels sont-ils ? d'abord, l'évolution de l'épidémie a toujours été une suite d'aléas, de mauvaises surprises, d'événements venant contredire ce qui était, la veille encore, perçu comme une vérité. Chaque mesure nouvelle est un choix difficile, mais nécessaire.

de prématurée et de dangereuse, mais elle s'est révélée efficace, juste et adaptée. Elle a été saluée à l'époque comme un modèle de déconfinement, que vous avez conduit, monsieur le Premier ministre. On nous a reproché ensuite,

cela n'a pas empêché l'Allemagne d'avoir une forte contamination. Confiner préventivement n'est donc pas la bonne solution. Il y a ceux qui auraient voulu, au contraire, laisser la France sans coercition, sans obstacle, dans une irresponsabilité que nous retrouvons parfois dans certains comportements.

Certains s'adonnent à des comparaisons hasardeuses avec d'autres pays, les bonnes mesures étant apparemment souvent prises ailleurs. La fascination pour l'étranger qui sévit aujourd'hui me surprendra toujours ! Probablement oublient-ils de mentionner

le Gouvernement ne prend pas de demi-mesures, il prend des mesures appropriées, graduées, pour faire face à l'explosion virale actuelle, et qui permettront de passer le pic dans quelques jours puis, dans quelques semaines, de revenir, grâce à la vaccination, à une vie presque normale.

Au moment de prendre une décision, aujourd'hui, on peut toujours contester toutes les mesures et, si j'en crois ce que disait ce matin un leader de l'opposition, il ne faut fermer ni les écoles ni les commerces. Mais alors, que faut-il faire face à cette situation explosive ?

d'abord, celle d'un Président de la République qui décide, comme si la V République avait atteint son plafond de verre en ces instants dramatiques ; celle, ensuite, d'un exécutif qui parle des « choix collectifs que nous avons faits Je vous le demande : quel choix collectif a été fait ? Le confinement, le déconfinement, le reconfinement, le confinement limité, la fermeture des commerces, le couvre-feu à dix-huit heures, à le conseil de défense ? Je crains, monsieur le Premier ministre, que nous n'ayons pas la même définition de ce qu'est un choix collectif dans une démocratie parlementaire. Une république moderne, comme la réclamait Pierre Mendès France en son temps, aurait nécessité que le débat parlementaire ait lieu avant l'allocution du Président de la République et que l'ensemble du corps législatif soit étroitement associé à toutes les décisions prises depuis maintenant un an. an. Depuis un an, c'est- hélas ! -le même schéma qui se reproduit sans qu'aucune leçon ait été retenue. Je constate que le Président de la République a demandé aux soignants un effort pour augmenter nos capacités de réanimation, mais ce qui est nécessaire, avant tout, c'est de disposer de plus de main-d'oeuvre et de moyens. Le Président s'est voulu rassurant, mais le constat est tout autre : l'épidémie a bondi, la vaccination, si elle est effective, est encore trop lente et nous payons tous le pari d'avoir privilégié temporairement l'économie, au risque d'un rebond fulgurant de la contamination. Je le dis sans ambiguïté il n'y a aucune intention pour notre part de soulever des polémiques inutiles, mais nous avons l'impression, avec regret, que l'ensemble des mesures prononcées hier auraient pu, et auraient dû, être prises en amont et que nous avons perdu un temps précieux. Sur ces mesures, je crois que nous pouvons tous partager l'objectif initial qui était de maintenir les écoles ouvertes. Maintenir ce lien entre l'école de la République et ses enfants était nécessaire, car on connaît les conséquences désastreuses d'un éloignement prolongé de l'école pour les élèves, notamment pour les plus défavorisés d'entre eux. Toutefois, si le virus ne circule pas plus à l'école qu'ailleurs, il n'y circule pas moins non plus, aussi, la fermeture annoncée était devenue inévitable. Face à cela, la simple annonce d'un calendrier de réouverture est insuffisante. Oui, vous avez annoncé le droit au chômage partiel pour l'ensemble des Français qui ne pourraient pas télétravailler, et ils sont nombreux, notamment dans les territoires ruraux. autant qu'il soit aisé de télétravailler avec des enfants à la maison ? Il faut aller plus loin en proposant des alternatives de garde, en prenant plus largement en compte les 8 millions de familles monoparentales de notre pays. Il faut, enfin, se servir de ces trois semaines de fermeture pour vacciner prioritairement les professeurs et les encadrants, ce qui permettra de concilier une réouverture rapide des classes et la protection sanitaire que nous devons à nos équipes éducatives. Sur la vaccination, toujours, on ne peut que souscrire au « Vacciner, vacciner, vacciner » et à la volonté de voir l'ensemble de la population vaccinée au plus tôt. là encore, on ne peut que regretter les atermoiements concernant la stratégie vaccinale. Atermoiements, d'abord, sur la commande européenne, plus que timide. Atermoiements, ensuite, sur le rythme de vaccination des plus âgés et des patients à risque. Atermoiements, enfin, quant à l'utilisation du vaccin AstraZeneca

même si nous sommes des Européens convaincus, il nous faut militer pour la levée des brevets concernant les vaccins et adapter notre appareil productif afin d'avoir la maîtrise de notre destin vaccinal. En somme, il nous faut agir plutôt que réagir pour atteindre nos objectifs de sortie de crise.

D'abord, dans les zones rurales, nombre de commerces et de services publics ou même de santé ne se situent pas dans un tel cercle, ce qui mettra automatiquement nombre de nos concitoyens hors la loi. Ensuite, comment vérifier une adresse lorsque celle-ci n'est pas la même que celle du papier d'identité ? Et lorsque l'adresse est la bonne, comment être sûr que le cercle des dix kilomètres est bien respecté ? Les agents de police et les gendarmes ne sont pas dotés de décamètres

c'est un débat préalable au Parlement, car c'est bien notre rôle de voter la loi et de contrôler votre action, conformément à l'article 24 de notre Constitution. Ce qui a manqué aussi, c'est la confiance dans les élus locaux, qui, souvent, sont les plus à même de prendre des décisions pour leur territoire. Mettons-nous à la place du maire de Cahors, de Tarbes ou de Mende, qui voient les décisions arriver d'en haut et subissent du jour au lendemain la fermeture de leurs commerces non essentiels sans avoir été consultés. Ce qui manque, au fond, c'est la confiance de nos concitoyens, des élus des territoires et de la majorité des membres du RDSE, dont vous connaissez pourtant l'attachement à nos institutions et la volonté de placer l'intérêt du pays au-delà de toute querelle partisane. L'unité aurait été de mise, ainsi que l'image d'une nation rassemblée face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Hélas, monsieur le Premier ministre, l'unité nationale ne se décrète pas : elle se construit. Aussi, vous comprendrez que notre groupe,

ne tenait pas aujourd'hui à un fil, si la vie sociale et économique du pays n'était pas bouleversée, le débat auquel vous nous convoquez aujourd'hui s'apparenterait à une mauvaise blague. Une nouvelle fois, le Président de la République a présenté seul, hier, des mesures pour lutter contre la pandémie, dont il a décidé seul, accompagné par le seul Conseil de défense. Le Parlement est donc définitivement perçu comme une chambre d'enregistrement, écartée progressivement depuis le début de la crise, et aujourd'hui, définitivement mise sur la touche. Nous sommes donc convoqués aujourd'hui pour vous écouter nous expliquer les décisions présidentielles, au cas où nous n'aurions pas bien compris. De surcroît, vous nous demandez de voter sur des propositions, d'une part, qui n'ont absolument pas été débattues préalablement, et, d'autre part, dont nous ignorons les motivations. En clair, nous ne savons pas pourquoi Emmanuel Macron a décidé certaines mesures qu'il rejetait quelques jours plus tôt, et pourquoi il en a écarté d'autres. Dès le début de la crise, le 19 mars 2020, nous avons alerté, ici même, au Sénat, sur le risque de dérive autoritaire que comportait l'état d'urgence sanitaire. Depuis des mois, nous demandons de renoncer à cet état d'exception qui met le couvercle sur la démocratie. Rappelez-vous, mes chers collègues, de la dernière prorogation : nous avons rappelé que l'état d'urgence n'était plus une justification et que la gravité de la situation exigeait de rendre au Parlement sa capacité permanente de décision. La représentation nationale, c'est la représentation du peuple, monsieur le Premier ministre. Le Parlement, c'est cela, et non un aréopage de gens inutiles, comme au temps du Conseil des M. Macron et vous-même renvoyez à l'opinion publique cette conception qui serait la vôtre du Parlement. Le mépris du Parlement est patent, et nous tenons à exprimer solennellement notre désaccord profond avec cette pratique institutionnelle. C'est même de la colère, monsieur le Premier ministre, car car nous constatons la mise en pratique de la volonté jupitérienne d'écarter le Parlement de sa route, alors que la révision constitutionnelle préparée par le chef de l'État n'a pu être imposée ni ici ni au pays. Cette dérive autocratique que beaucoup ont soulignée et dénoncée dès les premières heures du quinquennat prend une dimension inquiétante aujourd'hui, le Président de la République écartant tout de son chemin : Parlement, Conseil des ministres, puisque le Conseil de défense, détourné de son objet initial fixé par l'article 15 de la Constitution relatif au rôle de chef des armées du Président le supplée, et même le Conseil scientifique, puisque Emmanuel Macron, si l'on en croit les éloges de M. Blanquer, détient la connaissance, voire la science infuse en matière épidémiologique. L'exercice solitaire du pouvoir n'est jamais une bonne chose pour la démocratie ; en temps de crise, cela peut générer des drames. La reprise en main par le Parlement, par le collectif, par la démocratie devient une nécessité absolue. Hier soir, M. Macron nous a donc présenté ses choix : nouveau changement de pied avec la fermeture, brève pour l'instant, des établissements scolaires et l'abandon de la stratégie territoriale. On aura d'ailleurs noté cette étonnante initiative, au nom de la « respiration », d'autoriser la circulation dans tout le pays jusqu'au 5 avril, pour permettre sans doute aux propriétaires de résidences secondaires en particulier, de passer trois semaines ou le mois à venir au vert.

Monsieur le Premier ministre, le 29 janvier, lorsqu'a été prise la décision de ne pas reconfiner et de préférer des mesures de freinage, qui ont échoué, vous saviez que le variant anglais pouvait avoir des effets dévastateurs dans notre pays. médicale (Inserm) a mis en ligne une modélisation estimant que le variant anglais « deviendrait dominant entre fin février et mi-mars ». L'Inserm avait également annoncé le niveau d'hospitalisation auquel nous allons parvenir dans les jours à venir. Nous avons noté le scepticisme, au sein même du Gouvernement, concernant les annonces de Boris Johnson le 22 janvier sur un variant potentiellement plus mortel. une étude incontestée affirmait que ce variant anglais était « 64 % plus mortel ». M. Macron le savait, vous saviez ; pourtant, vous avez attendu d'être dos au mur, celui de la saturation des services de réanimation,

Mais il y a une vérité que M. Macron a dissimulée hier en demandant encore plus d'efforts aux soignants : c'est cette saturation et les tris déjà engagés, puisque, ne jouons pas sur les mots, déprogrammer des opérations, c'est bien trier des malades

Monsieur le Premier ministre, je vous ai interrogé ici même, au Sénat, il y a quinze jours sur la promesse non tenue depuis un an d'ouverture de ces lits de réanimation. Vous avez indiqué que de tels lits ne pouvaient se commander chez Ikea ni être créés en un claquement de doigts. Vous ne pouviez pas ; M. Macron l'a fait. Qu'en pensez-vous ? Le Président cherche-t-il à faire oublier qu'avec vous il poursuit, contrairement à ses dires depuis un an, la fermeture des lits ? Ce qui a été annoncé hier, c'est l'absence totale d'anticipation, soulignée par la Cour des comptes, en matière de réanimation. vous le dire, monsieur le Premier ministre, mais votre gouvernement est resté les deux pieds dans le même sabot en la matière, engoncé dans le dogme libéral d'économie de la dépense publique. Les conséquences sont aujourd'hui dramatiques. Le « quoi qu'il en coûte » n'a pas été appliqué pour l'hôpital. Monsieur le Premier ministre, l'espoir, c'est le vaccin. Là aussi, vous avez failli et, avec vous, le système tout entier, cette fameuse loi du marché que dénonçait Emmanuel Macron dans son discours du 12 mars 2020. Le retard mortifère pris en matière de vaccination trouve son origine dans le fléau de la concurrence, du profit, des gains réalisés grâce à la maladie. Les petits mensonges et autres travestissements de la vérité, les vaccinodromes que l'on moque puis que l'on convoque en urgence, les élus municipaux que l'on critique, que l'on bride mais qui sauvent la situation : tout cela n'aurait pas eu lieu si le vaccin avait été promu comme un bien commun, sorti des logiques capitalistes pour servir l'intérêt général, sans autre profit que la protection de l'humanité. Pourquoi la France n'agit-elle pas pour la levée des brevets ? Pouvez-vous nous répondre, monsieur le Premier ministre ? Quelle est la boussole du Président : la santé de nos compatriotes ou le sauvetage d'une économie mondialisée en crise profonde ? La question mérite d'être posée. J'en viens, enfin, à l'école. Oui, maintenir les écoles ouvertes est un souhait largement partagé, et nous le partageons ; mais à quel prix ? Donnez-nous les éléments : combien de vies ont-elles été perdues ? Chacun ici a un proche ou un ami malade ou décédé du fait du retard pris pour limiter l'expansion du variant anglais. Les jours et les semaines à venir apporteront cette réponse. Monsieur le Premier ministre, ce débat- je l'ai dit d'emblée -ne respecte pas le Parlement. Nous devrions débattre des mesures à prendre, mais elles sont déjà prises. C'est la confiance que vous devriez aujourd'hui demander au Parlement et, croyez-moi, nous ne vous l'aurions pas accordée tant la gestion de cette épidémie est contraire aux intérêts de notre pays, de notre peuple. avec la quasi-totalité des groupes politiques du Parlement, nous avons décidé, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote sur votre déclaration, car cette consultation n'est pas respectueuse de la Constitution et, qui plus est, elle est marquée, monsieur le Premier ministre, d'une certaine hypocrisie. La parole est

Le Président de la République a souhaité que les enseignants, eu égard au fait que les classes sont restées ouvertes beaucoup plus longtemps que dans les pays qui nous entourent, puissent être vaccinés rapidement. Il a également évoqué les forces de l'ordre,

mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne manqueriez pas de nous en faire reproche d'ici à quelques semaines, considérant que nous aurions joué avec la santé des Français. Depuis le début de cette crise, le leitmotiv est qu'il faut aller vite- vous avez raison -, qu'il faut aller fort, qu'il faut refuser tous les blocages, tous les obstacles quand ils sont inutiles, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.

ne se sont pas avérées gagnantes. Monsieur le président Retailleau, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler les débats que nous avons eus sur un médicament dont on sait aujourd'hui qu'il ne fonctionne pas. Très bien ! J'ai même été rendu coupable de ne pas vouloir le prescrire comme des bonbons à tous les Français.

intense. Il y a un an, j'avais demandé l'activation du plan blanc dans tous les hôpitaux, en exigeant la déprogrammation de tous les actes dans toute la France pour que nous soyons prêts, parce que nous ne savions pas à quelle vitesse monterait la vague. Aujourd'hui, nous savons à quelle vitesse monte la vague : entre 50 et 100 patients sont admis en réanimation chaque jour.

n'a empêché le variant de monter ni en Allemagne, ni en Italie, ni dans les autres pays qui ont confiné pendant des semaines et des mois. Aujourd'hui, nous pouvons constater que nous avons gagné du temps, du temps de liberté, certes sous contrainte et avec un couvre-feu, mais du temps de liberté quand même. Les commerces et les écoles sont restés ouverts en France beaucoup plus longtemps qu'à l'étranger.

que, si avec beaucoup de ministres de mon Gouvernement, je suis ici, devant vous, cet après-midi, c'est précisément parce que je respecte beaucoup le Parlement et le Sénat.

ce serait le priver des droits et des prérogatives qu'il tient de notre Constitution et des institutions de la V République.

En application de l'article 34 de la Constitution, tout ce qui dans la gestion de cette crise sanitaire relève du Parlement est soumis au Parlement. Comme je l'ai dit ce matin devant l'Assemblée nationale,

-sur des prérogatives du pouvoir exécutif. De vous à moi, je ne suis pas certain que le général de Gaulle, auquel je voue un immense respect, n'aurait pas trouvé iconoclaste qu'un gouvernement vînt demander au Parlement l'approbation de dispositions relevant de son autorité. C'est pourtant ce que nous faisons.

Vous avez sans doute observé comme moi qu'ils ne se privent pas de s'en saisir pour commenter et critiquer- c'est leur droit élémentaire en démocratie -l'action des pouvoirs publics et du Gouvernement. Chaque fois que le Parlement nous pose des questions, nous répondons. Chaque fois que le Parlement, dans le cadre des pouvoirs légitimes de contrôle qui sont les siens, qui sont les siens, nous interroge, nous répondons. Telle est d'ailleurs l'instruction que je donne quotidiennement aux ministres. En ce sens,

en considération de la représentation nationale, je viens expliquer les tenants, les motivations et le contenu des mesures difficiles que le Gouvernement s'apprête à prendre en vertu des pouvoirs que la Constitution démocratique de notre pays lui a attribués. Rien de plus, mais rien de moins. Je vous le dis sans le commenter, car c'est votre choix : prendre part à ce vote, dans le sens qu'en votre âme et conscience vous auriez souhaité lui donner,

et elle va, ici comme ailleurs, plus vite que la vaccination. Elle nous oblige à prendre des mesures complémentaires sur lesquelles je suis venu vous rendre des comptes. Mais soyons clairs ! Le

parmi d'autres, est extrêmement illustratif. Certains médecins expliquent qu'il faut fermer les écoles, quand leurs collègues pédiatres et non moins médecins, me semble-t-il, recommandent l'inverse.

Il va falloir nous serrer les coudes. Je ne le dis pas forcément à titre politique, car je ne suis pas naïf. Je le dis pour notre pays, pour faire face à cette nouvelle épreuve. Je vous trouve toutes et tous, et je vous le dis tel que je le pense, particulièrement sévères. C'est votre droit.

qu'on pourrait trouver plus de doses qu'il n'y en a, cela n'est ni raisonnable ni responsable. Notre devoir, en revanche, c'est de vacciner autant que possible dès que toutes les doses seront là. Le devoir de l'Europe, c'est de faire respecter les contrats qu'ont souscrits les industriels et les laboratoires. Croyez bien que nous nous y employons avec la dernière énergie ! Mesdames, messieurs les sénateurs, le système de santé est très éprouvé. Je le redis à ceux qui se sont exprimés : là non plus, ne faisons pas croire qu'on peut créer des lits de réanimation en un an

La séance est suspendue.

qu'auparavant la confiance et les marges de manoeuvre sur lesquelles nous nous étions engagés dans le cadre du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, ce sont des sommes d'un montant sans précédent qui ont été mises sur la table, des revalorisations ambitieuses depuis septembre et des investissements pour l'ensemble du système de santé,

Elles ont été étendues aux personnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux rattachés aux hôpitaux publics par un accord, le 16 février dernier. Des négociations se poursuivent pour rendre ces métiers du public plus attractifs. Il n'y aura pas d'oubliés du Ségur Au-delà de ces revalorisations salariales, attendues depuis longtemps, par-delà les âges et les alternances, le Ségur de la santé a permis de partager un diagnostic d'ampleur. Qu'il s'agisse d'investissements pour regarder l'avenir avec confiance, qu'il s'agisse de gouvernance pour assurer une juste participation de ceux qui soignent, qu'il s'agisse de l'élargissement des compétences des professionnels de santé, nous n'avons éludé aucun sujet. Certaines des avancées introduites par la Haute Assemblée ont été conservées par l'Assemblée nationale.

a été présentée en conseil des ministres le 17 mars dernier. Les commissions médicales de groupements seront demain des instances décisionnelles dans la vie de ces établissements. Par conséquent, les missions des commissions médicales d'établissement et de groupement, et leur président sont ainsi revus, conformément aux recommandations du rapport du professeur Claris, qui ont fixé le cap que nous suivons. Par ailleurs, le Ségur a préconisé la réhabilitation « du rôle et de la place du service au sein de l'hôpital », en reprenant notamment une préconisation du rapport Claris. Cette proposition de loi répond également, vous le savez, à la revendication ancienne des acteurs locaux, qui souhaitent disposer d'une plus grande liberté d'organisation interne, s'agissant par exemple des établissements de santé. La crise a montré, et nous démontre encore, que les collectifs de soins savent s'adapter, s'organiser et surmonter des situations extrêmement sensibles, sans attendre pour cela un accord, une validation ou un feu vert venu d'en haut.

Nous devons continuer de progresser en matière de démocratie hospitalière. Ce texte propose justement de faire siéger au directoire des établissements publics hospitaliers un représentant des personnels non médicaux, un représentant des étudiants en santé et un représentant des usagers dont nous avons à apprendre. C'est une liberté donnée aux acteurs et nous y tenons, car c'est encore un gage de confiance. Par ailleurs, le Gouvernement s'est engagé fortement dans la lutte contre le mercenariat de l'intérim médical, qui désorganise l'offre de soins dans nos territoires et met à mal les finances de nos hôpitaux. Vous aviez eu un débat intéressant, en première lecture, qui a démontré les limites des dispositions actuelles et la nécessité d'aller plus loin dans le contrôle de l'intérim pour mettre fin aux dérives. Le texte ainsi rédigé permet une bonne fois pour toutes de rendre effectif le plafond réglementaire de l'intérim médical en obligeant le comptable public à rejeter tout paiement au-delà de ce plafond. Cette proposition de loi renforce également un certain nombre de mouvements nés cet été avec le Ségur de la santé. L'un de ces mouvements est l'extension du champ de compétences de certaines professions. Je pense en particulier aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux orthophonistes et aux ergothérapeutes. Ouvrir le champ des actes ouverts à ces professions, c'est faire le choix de la confiance et de l'efficacité. Nous faisons le pari que notre système de santé ne sera en mesure de relever les défis auxquels il fait face qu'en rompant avec les querelles de chapelles et les prés carrés dans lesquels certains souhaiteraient nous enfermer. De la même manière, nous avons élargi l'étendue du rapport sur les protocoles de coopération et pratiques avancées à la question spécifique de l'accès à des pratiques avancées aux infirmiers spécialisés, notamment aux infirmiers anesthésistes, afin de reconnaître leurs compétences. J'ai tenu à revenir sur les principaux axes de cette proposition de loi, car ils constituent autant d'évolutions attendues par les acteurs et pour notre système de santé.

Alors que notre système de santé est soumis à une pression inédite, le texte, à ce moment de nos discussions, laisse un goût d'inachevé : sans vraiment tirer les enseignements de la crise, il peine à répondre aux vives attentes exprimées lors du Ségur de la santé faire confiance et simplifier. En raison d'un trop grand nombre de divergences entre l'approche du Sénat et celle de l'Assemblée nationale, à l'origine de cette initiative, la commission mixte paritaire réunie le 2 mars dernier n'est pas parvenue à établir un texte commun. La poursuite de la navette a confirmé certains apports de la Haute Assemblée l'élargissement de la vaccination aux biologistes, la prescription d'aides techniques par les ergothérapeutes, la désignation d'une sage-femme référente dans le parcours de grossesse ou celle de référents handicap dans les hôpitaux. Nous avons aussi convergé pour rejeter le bénévolat individuel dans le contexte sensible des établissements de santé ou pour autoriser les professionnels hospitaliers des établissements de santé privés à intérêt collectif (Espic) à maintenir des dépassements d'honoraires sans menacer l'accès aux soins. De même, sur la gouvernance hospitalière, les députés ont retenu la clarification opérée par le Sénat entre la fonction de chef de service et celle de chef de pôle, une meilleure association de la commission des soins infirmiers à la conception du projet d'établissement. Cependant, si nous saluons ces convergences ponctuelles, trop de dispositions formant le coeur de ce texte nous opposent, sans que la navette ait permis à ce stade

de deux des onze ordonnances promises par la loi Santé sur les GHT et sur l'attractivité des carrières hospitalières que nous devons le rejet systématique, et quelque peu contraint, par l'Assemblée nationale des dispositions que nous avions introduites en première lecture. C'est là une curieuse façon de légiférer, qui fait d'un projet d'ordonnance encore en gestation le censeur politique de nos amendements sur des dispositions connexes. Tel a donc été le sort de nos articles, qui prévoyaient un maillage plus pertinent et mieux intégré de l'offre de soins, en rendant notamment obligatoire l'élaboration du projet territorial de santé, afin que la structuration de l'offre suive une trajectoire réellement ascendante. De la même façon, et malgré la volonté revendiquée dans le texte initial de traduire par voie législative les recommandations issues des concertations du Ségur de la santé, la demande exprimée par les personnels paramédicaux d'une participation accrue à la direction de l'établissement et d'une plus grande représentativité du président de la commission des soins infirmiers, que nous avions satisfaite en première lecture, n'a pas été acceptée par l'Assemblée nationale. Nous avons en revanche été davantage surpris que l'Assemblée nationale, en ressuscitant l'article 8, que nous avions préalablement supprimé, charge la commission des affaires sociales du Sénat de désigner, à partir de critères non définis, la sénatrice ou le sénateur qui aura qualité pour siéger au conseil de surveillance de l'établissement principal des établissements publics de santé. Cette disposition nous semble inapplicable en l'état et, sur la forme, assez discourtoise. Nous aurons à coeur de la supprimer dès que possible. Enfin, madame la ministre, je veux rappeler solennellement devant vous notre position au sujet de la lutte contre l'intérim médical. Animés de la même intention que vous, nous avions néanmoins tenté de vous alerter sur les faux espoirs que suscite l'idée, juridiquement bancale, d'un contrôle de légalité de la dépense d'intérim par le comptable public opéré à l'issue de l'engagement de cette dernière. Le circuit de la dépense publique, qui oblige ses ordonnateurs à l'égard des prestataires qu'ils sollicitent, ne permet pas que le contrôle d'opportunité de la dépense intervienne au moment de son paiement. Les intérimaires ayant signé, le plus souvent avec des directeurs d'hôpitaux contraints, des conventions de prestations parfaitement légales contesteraient ce défaut de paiement devant les tribunaux administratifs et remporteraient leur contentieux. L'Assemblée nationale a considéré que le recours aux instruments budgétaires ordinaires de l'hôpital, dont on déplore souvent l'excès de détails, n'était pour l'occasion pas assez précis pour détecter en amont un recours abusif à l'intérim.

irrégulière, dès le stade de l'engagement, et neutralise le risque de contentieux ultérieur. L'avenir seul dira si nos craintes étaient justifiées et si la solution que vous proposez est opérante. Permettez-moi, mes chers collègues, de conclure ce propos par un sujet qui, bien que ne figurant pas explicitement dans la proposition de loi, ne peut être passé sous silence, alors que nous débattons de l'avenir de l'hôpital public. Je veux évoquer les craintes nombreuses et légitimes qu'expriment en ce moment, à l'approche des épreuves de sélection pour l'entrée en deuxième année, les étudiants en santé de première année, qui achèvent cette première étape de leur parcours en faisant face, pour un nombre de places identique, aux anciens étudiants de la Paces de l'an dernier admis au redoublement. Le prédécesseur de l'actuel ministre de la santé avait fort bien anticipé ce problème, en promettant lors du vote de la loi Santé seule année, un pourcentage supplémentaire d'étudiants admis en deuxième année soit spécifiquement dédié à la gestion de ces redoublants, afin de ne pas créer d'inégalités au détriment des étudiants primants. Les chiffres progressivement arrêtés par les différentes universités, dont la transparence s'est malheureusement dégradée depuis la mise en place du, confirment que cet engagement ne sera malheureusement pas respecté.

le Président de la République a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de covid-19. Aujourd'hui, le Sénat débute l'examen en nouvelle lecture de la proposition de loi visant à améliorer notre système de santé. Or nous savons toutes et tous que notre système de santé souffre, plus que jamais avec cette pandémie, d'un manque de lits, de personnels et de services surchargés. Nous savons pertinemment que les personnels soignants, qui sont en première ligne, sont épuisés. La tension est tellement forte que bon nombre de médecins nous alertent sur le risque d'un tri des patients dans les services de réanimation, mais également sur les déprogrammations d'interventions chirurgicales, entraînant des pertes de chance. D'ailleurs, les nouvelles restrictions annoncées par le Président de la République sont en partie liées à l'insuffisance de nos capacités hospitalières, ce qu'il n'a pas caché. Notre groupe ne cesse de dénoncer les politiques menées depuis plus de vingt ans, qui, de coupes budgétaires en coupes budgétaires, sont responsables de l'état de nos hôpitaux publics et de l'affaiblissement de notre système de santé. Cette proposition de loi n'est pas à la hauteur des enjeux : elle est déconnectée de la réalité des hôpitaux et n'est pas de nature à redresser la barre. Pis, certaines mesures vont encore aggraver la situation. Ainsi, en renforçant l'autonomie des hôpitaux et des groupements hospitaliers de territoire, ce texte affaiblit encore davantage le service public national de santé. On le voit déjà dans les projets en cours. Pour ne prendre qu'un exemple, la création programmée à Saint-Ouen d'un hôpital-cathédrale pour remplacer les hôpitaux Bichat et Beaujon va entraîner la suppression de près de 400 lits et de 1 200 emplois. Comment justifier que la modernisation indispensable de ces hôpitaux provoque une réduction des capacités d'hospitalisation dans une zone qui souffre déjà d'un manque de structures hospitalières ? Ce que demande la coordination composée de personnels, de syndicalistes, d'élus, de patients, d'habitantes et d'habitants du secteur, c'est non seulement de moderniser Bichat et Beaujon,

Aujourd'hui, à l'école, on observe une pénurie de médecins et de psychologues scolaires. Il faut donc embaucher, revaloriser ces professions et non modifier leurs missions. Deuxièmement, concernant la demande ancienne des orthophonistes visant à autoriser l'accès direct aux soins orthophoniques, afin de mieux orienter un certain nombre de patients et de fluidifier leur parcours de soins, nous regrettons les reculs du Gouvernement face à la pression de certaines corporations, qui a entraîné la suppression de l'amendement adopté par le Sénat dans un très large consensus. Madame la ministre, je vous alerte sur ce point. point. Troisièmement, je veux redire ici qu'il y a urgence à inclure dans les objectifs du projet social des hôpitaux la lutte contre les comportements sexistes, racistes et homophobes.

dans neuf cas sur dix, le harceleur était un supérieur. Beaucoup de manques, des propositions qui confortent les politiques menées jusqu'à présent : autant de raisons pour nous opposer à cette proposition de loi en nouvelle lecture comme en première lecture. La parole

Je suis donc très ennuyée par une proposition de loi dont la rédaction ne semble pas convenir à de nombreuses professions. C'est particulièrement problématique. Avec les membres de mon groupe, nous avions approuvé et salué les mesures budgétaires du Ségur, tout en soulignant que certains Aujourd'hui, cette proposition de loi, qui se voulait la traduction des mesures non budgétaires du Ségur de la santé, n'atteint que très partiellement cet objectif. Je retiens néanmoins de ce texte les avancées bienvenues concernant la profession de sage-femme. Le chapitre II lui est majoritairement consacré. Il prévoit notamment la possibilité pour la patiente de désigner une sage-femme référente, afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin. Il sera aussi désormais possible pour une sage-femme d'adresser ses patientes à un médecin spécialiste, sans pénaliser ces dernières pour ce qui est du remboursement des soins par l'assurance maladie. Il s'agit d'une Il s'agit d'une mesure de simplification du parcours de santé là encore bienvenue. Tel est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi. Je rappelle enfin le point de vigilance que j'avais soulevé en première lecture nous ne pouvons étendre indéfiniment le champ d'intervention des professionnels sans améliorer leur statut, qui est actuellement hybride, puisqu'il est médical devant la loi, mais souvent paramédical pour l'administration.

l'heure est aux mesures concrètes. Elles demandent notamment une augmentation des effectifs, la reconnaissance de leur statut de profession médicale à l'hôpital, un alignement des salaires sur les autres professionnels de santé, ainsi que l'ouverture de négociations conventionnelles dans le cadre du rapport des 1 000 Je souhaite que la mission de l'IGAS, qui devrait remettre ses conclusions d'ici à l'été, puisse aboutir à des mesures à la hauteur des enjeux lors du prochain projet Je ne m'étendrai pas davantage sur le fond du texte. Je vous redis mon malaise et ma perplexité, après toutes les auditions et le travail mené sur cette proposition de loi. Je regrette que le Sénat et l'Assemblée nationale n'aient pu s'entendre. De nombreux points de divergence nous séparent. Aussi, je ne vois pas ce qui peut nous réunir au-delà de quelques articles consensuels que le Sénat a améliorés. Je partage l'analyse de notre rapporteur Alain Milon Milon : « sur le coeur des dispositions, l'Assemblée nationale a rétabli, pour l'essentiel, son texte de première lecture », notamment en matière de gouvernance hospitalière, alors que le Sénat avait adopté des propositions constructives sur des points concrets de cette évolution. Dans ces conditions, poursuivre le débat n'aurait pas tellement de sens et risquerait en définitive de créer de faux espoirs chez les professionnels de santé. Aussi, les sénateurs du groupe Union Centriste prennent acte de l'échec de la commission mixte paritaire et voteront la motion tendant à opposer la question préalable.

proposition de loi dans un contexte marqué par la crise que nous connaissons. Il y a un an, les Françaises et les Français applaudissaient spontanément le personnel soignant. Après une année très difficile, un dévouement sans précédent de ces personnels, le décès de beaucoup d'entre eux, tous avaient imaginé une prise de conscience collective et un appui ferme et unanime des pouvoirs publics.

Cette proposition de loi apparaît plus que jamais en décalage avec les besoins matériels et humains dont notre système de soins a besoin. C'est la raison pour laquelle l'écrasante majorité des syndicats et des associations de professionnels de santé s'est positionnée contre son adoption. Vous avez fait le choix de légiférer dans une certaine forme de précipitation. Malgré d'importantes contributions du Sénat, l'Assemblée nationale a, pour l'essentiel, de loi avait pour ambition de réaffirmer le rôle des services et du chef de service dans la gouvernance de l'hôpital. Nous pensons en effet qu'ils constituent une unité pertinente dans la prise de décision, dans l'organisation et la mise en oeuvre de l'offre de soins, et que les réformes successives de l'hôpital les ont trop éloignés des instances décisionnelles. Mais, au fond, ce texte ne procède ni à un réel changement de cap ni à une nouvelle répartition des compétences entre les pôles d'activité et les services qu'attendent pourtant les personnels hospitaliers.

Par exemple, vous n'avez pas tiré les enseignements du printemps dernier lorsque l'hôpital, malgré la surcharge extrême, fonctionnait mieux, car l'administration était au service des soignants, et non dans la complication et la limitation permanente de leur action. Confiance et simplification », dites-vous, quand le 17 mars dernier, à l'issue du conseil des ministres, le Président de la République a signé deux ordonnances déclinant les dispositions de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. L'une de ces ordonnances est « relative aux groupements hospitaliers de territoire et à la médicalisation des décisions à l'hôpital », quand l'autre vise « à favoriser l'attractivité des carrières médicales hospitalières ». Sur la forme, vous ne respectez pas le principe de l'ordonnance. En juillet 2019, le Parlement vous donnait sa confiance pour légiférer de la sorte, afin de vous donner le temps d'un travail rigoureux associant l'ensemble des représentants des professions concernées. À l'arrivée, comment pouvez-vous estimer que les concertations ont été menées dans de bonnes conditions, alors qu'il en résulte un rejet massif des organisations syndicales ?

pour la première, à un vote unanimement défavorable de l'ensemble des représentants des praticiens et, pour la seconde, à un vote majoritairement défavorable de cette représentation ». Voilà comment les premiers concernés jugent cette loi.

ne sont toujours pas tirées. En vérité, soignants comme parlementaires, nous attendons une loi Santé à la hauteur de l'engagement de nos professionnels de santé, de santé, des transformations nécessaires du système de soins. Nous en sommes tellement loin que la poursuite de ce débat ne nous semble pas utile. C'est la raison pour laquelle nous voterons la motion tendant à opposer la question préalable. La parole

Je regrette, comme beaucoup d'entre nous, l'échec de la commission mixte paritaire le 2 mars dernier et la suppression par l'Assemblée nationale de la plupart des mesures adoptées par le Sénat. Les désaccords portent essentiellement sur trois points : les protocoles de coopération et la création d'une profession médicale intermédiaire, les moyens de lutter contre les dérives de l'intérim médical et la gouvernance hospitalière. L'amendement de notre collègue Alain Marc visant à étendre le dispositif d'exercice en pratique avancée aux infirmiers anesthésistes a été supprimé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. La disposition proposée par Franck Menonville tendant à renforcer le rôle des élus au sein du conseil de surveillance des établissements de santé a également été supprimée. D'autres mesures importantes ont connu un sort similaire. Je pense notamment à l'autorisation de primoprescription et à la délivrance du traitement de prévention du VIH par les médecins de ville et les pharmaciens, que le Gouvernement a jugé prématurées. Lorsqu'il est question de la santé de nos concitoyens, je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour agir. La navette parlementaire a néanmoins contribué à enrichir le texte. La possibilité de désigner une sage-femme référente a été maintenue, ainsi que l'extension de l'acte de vaccination aux pharmaciens et aux biologistes. Les orthophonistes, les masseurs-kinésithérapeutes et les ergothérapeutes auront bientôt la possibilité d'adapter des prescriptions médicales. Ces mesures concrètes contribueront à faciliter le parcours de soins des patients. Je partage la réflexion de notre rapporteur, Alain Milon, sur l'article 1 instituant une nouvelle profession médicale. L'exercice en pratique avancée répond précisément à l'objectif d'ajouter un maillon supplémentaire dans l'offre de soins, sans pour autant la rendre plus complexe et, donc, moins accessible. En revanche, je suis favorable à certaines avancées plus volontaristes de l'Assemblée nationale en matière d'accès à la santé : le renouvellement des arrêts de travail de plus de quinze jours par par l'ensemble des sages-femmes, la prescription de traitements des IST aux partenaires, ainsi que leur autorisation à orienter leurs patientes vers la médecine spécialisée. outre, la création de la plateforme numérique d'accès au droit pour les personnes en situation de handicap est une disposition importante de cette proposition de loi. Mon collègue Daniel Chasseing avait proposé en séance publique d'étendre le bénéfice de cette plateforme aux personnes âgées dépendantes. L'examen du projet de loi Grand Âge sera l'occasion de réexaminer cette mesure. Le texte contient des avancées intéressantes. Conformément aux usages de notre groupe, nous avons choisi de ne pas voter la motion déposée par la commission, car nous souhaitons poursuivre les discussions et l'examen des amendements que nous avons déposés. La parole

lors de la première lecture, nous avions relevé la déception et les inquiétudes de la majorité des acteurs de santé quant à cette proposition de loi : le texte marquait une véritable incapacité à se saisir des enseignements de la crise sanitaire pointés lors du Ségur de la santé. santé. Sur le versant financier, malgré un début de rattrapage du décrochage des rémunérations, le Gouvernement n'en poursuit pas moins aujourd'hui les projets de fermeture de lits. De même, le versant dit « non financier » du Ségur témoigne d'un rendez-vous en grande partie manqué. Aujourd'hui même- ce n'est pas un poisson d'avril ! -, l'hôpital militaire Desgenettes de Lyon ferme ses urgences alors que son service de médecine, sous-employé, pouvait accueillir les patients covid ne nécessitant pas ou plus de réanimation, à deux pas de l'hôpital public Édouard-Herriot désormais saturé. La casse continue. Comme les acteurs de santé, nous avons apporté notre contribution pour que cette crise ouvre sur une rénovation profonde de notre système de santé. Au Sénat, le travail parlementaire avait permis de supprimer les articles unanimement contestés lors des auditions. Le groupe écologiste avait ainsi salué quelques avancées. Je pense bien sûr à la possibilité pour la femme enceinte de désigner une sage-femme référente et à l'accès direct aux soins d'orthophonie, défendu largement sur nos travées. La majorité des articles les plus contestés ont été rétablis par l'Assemblée nationale, notamment l'article relatif à la compétence de recrutement donnée à l'établissement support du GHT pour le compte des établissements parties. Ce rétablissement valide l'analyse et les craintes des acteurs locaux de santé. Ces derniers redoutent une intégration principalement au service d'une logique d'économies et non, malheureusement, pour construire une offre hospitalière efficiente maillant l'ensemble du territoire. Le bilan de la réforme de la gouvernance hospitalière reste bien pauvre. Ainsi, l'Assemblée nationale valide la suppression de la concertation interne préalable à la nomination du chef de service, demandée par la majorité sénatoriale, mais elle n'a pas l'audace d'expérimenter l'élection de ce même chef de service par ses pairs. L'article qui renforce la lutte contre le recours abusif à l'intérim, objectif qui fait l'unanimité, ne s'attaque nullement aux causes de ce phénomène. La pénurie dans certaines spécialités médicales, aggravée par le décrochage des rémunérations des praticiens hospitaliers- que certains préfèrent l'exercice en clinique privée -, explique le recours aux dépassements d'honoraires jusqu'au mode le plus dégradé, l'intérim, avec les abus Les injonctions paradoxales faites aux directeurs- continuité du service, refus du chantage ou fermeture des services -ne sauraient constituer la seule réponse, pour ne pas dire la défausse du Gouvernement.

Une telle impéritie, un tel passage en force nous conduisent à condamner la méthode en plus du fond : nous ne voyons plus, nous non plus, l'intérêt de poursuivre l'examen de ce texte. Le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires votera en conséquence la question préalable.

vrai des décisions en matière de politiques publiques. La confiance mutuelle des acteurs de la santé est le préalable nécessaire à toute simplification dans ce elle, est devenue un enjeu majeur pour permettre à chaque soignant d'effectuer sa mission au mieux et à chaque patient d'être soigné et remboursé efficacement. Pendant cette crise sanitaire, cette simplification a prouvé sa nécessité absolue : d'une part, pour désengorger les urgences ; d'autre part, pour permettre la continuité des soins habituels. À ce titre, l'élargissement de la télémédecine remboursée pour tous, quel que soit le département du médecin, a permis d'assurer l'accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées, comme mon département de l'Eure. J'ai d'ailleurs écrit il y a quelques jours à M. le ministre des solidarités et de la santé pour lui demander la pérennisation de cette simplification au-delà de la crise sanitaire. de loi dont nous débattons aujourd'hui constitue la traduction législative des mesures issues des conclusions du Ségur de la santé, pour la partie non budgétaire. Le texte a été enrichi lors de sa première lecture au Sénat, et je souhaite souligner le travail du rapporteur, Alain Milon, et de la commission des affaires sociales. introduites par le Sénat ont été conservées par l'Assemblée nationale. Je pense à l'ouverture du droit de vaccination aux pharmaciens et biologistes ou encore aux dépassements d'honoraires des professionnels libéraux en Espic.

du système d'information au sein des groupements hospitaliers de territoire ; et l'article 14 A, permettant la mise en place d'un référent handicap au sein de chaque établissement de santé.

Face à ces modifications, une motion tendant à opposer la question préalable a été déposée. Or il serait regrettable d'arrêter ici les échanges : ce texte contient des mesures essentielles, demandées par les soignants depuis des années. D'autres méritent sans doute encore un travail d'amélioration, mais elles ne justifient pas un tel rejet en bloc. Les demandes des professionnels de santé ont été entendues, avec notamment 754 millions d'euros supplémentaires engagés en faveur des urgences pour la période 2019-2022. Le rapport Claris et le Ségur de la santé ont permis de préciser ces demandes. Cette proposition de loi représente ainsi plusieurs avancées concrètes l'élargissement des protocoles locaux de coopération ; l'évolution du rôle des sages-femmes, qui pourront notamment prescrire des arrêts maladie et les prolonger ; l'élargissement du droit de prescription pour elles et les masseurs-kinésithérapeutes ; la réinstallation de la fonction de chef de service ; la lutte contre les dérives de l'intérim médical ; ou encore la prise en compte des étudiants en santé dans l'élaboration du projet social.

C'est un signal positif que nous leur adressons. Pour lutter contre les dérives de l'intérim, l'Assemblée nationale a rétabli le dispositif permettant aux directeurs généraux des ARS de déférer devant le tribunal administratif les contrats irréguliers tout en donnant des pouvoirs au comptable public. public. Certains considèrent qu'un tel dispositif peut mettre les directeurs d'établissement en difficulté. Nous pensons au contraire qu'il leur enlève une responsabilité et les protège. Un bilan d'étape sera nécessaire sur ce point, qu'il faudra évaluer avec prudence et pragmatisme. A également été rétablie l'intégration d'un projet managérial au projet d'établissement des établissements publics de santé ; nous sommes convaincus de son utilité. On ne saurait réduire la maîtrise des techniques managériales à des enjeux de rentabilité. Bien au contraire, elles permettent d'améliorer le fonctionnement des équipes et des services. Je salue le maintien par l'Assemblée nationale de plusieurs de nos propositions. Je pense notamment à l'extension des compétences des professions paramédicales : l'idée était d'étendre le champ de leurs prérogatives. Ainsi, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les masseurs-kinésithérapeutes ont vu leurs droits de prescription étendus. Je pense également à la possibilité donnée aux pharmacies à usage intérieur et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale d'effectuer certains actes de vaccination, propositions que le groupe du RDSE avait introduites. Néanmoins, nous déplorons la suppression de certains apports du Sénat, comme le déploiement de l'exercice en pratique avancée des infirmiers anesthésistes, que notre groupe a défendu. Nous aurions souhaité faire plus pour l'attractivité des métiers, parvenir à une équité entre secteurs public et privé d'intérêt collectif. Nous avions proposé à ce titre de permettre aux praticiens salariés d'un Espic de pratiquer des dépassements d'honoraires, dans la limite des dispositifs prévus par la convention médicale. À notre regret, cette possibilité n'a été retenue que pour les professionnels les pratiquant déjà au 24 juillet 2019, date de promulgation de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Ce choix risque d'avoir pour effet de créer une nouvelle inégalité, au sein des Espic cette fois-ci. À l'issue du Ségur, qui avait suscité beaucoup d'espoirs, force est de constater que le présent texte répond insuffisamment aux ambitions. Il vient tout de même compléter des mesures qui étaient attendues- il ne faut pas le nier -et contribue à la remédicalisation de la direction de l'hôpital.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la nouvelle lecture, en séance publique, de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Cette lecture devrait être assez rapide- sans préjuger, bien sûr, le résultat du vote de la motion tendant à opposer la question préalable. Après une commission mixte paritaire elle-même rapide, témoignant ainsi des profondes divergences qui opposent la chambre haute et la chambre basse, nous avions toutefois secrètement l'espoir que la majorité gouvernementale daigne conserver certains apports votés au Sénat. Dire que nous avons été déçus est un euphémisme, mais cela n'est rien à côté de la déception des professionnels de santé ; déception d'autant plus grande que leur engagement au service des patients est sans faille depuis le début de la pandémie.

sujet plus transversal et consensuel que la santé ? Pourtant, vous avez réussi à fédérer l'ensemble des groupes d'opposition des deux assemblées contre ce texte, pas toujours pour les mêmes raisons, mais avec un constat partagé : cette proposition de loi ne résout pas l'essentiel. Face au mécontentement croissant des professionnels de santé, il était devenu impératif d'agir avec détermination afin de répondre à cette détresse, révélée au grand jour par la pandémie de la covid-19. Un calendrier particulièrement serré ne vous a pas laissé le temps de préparation nécessaire à l'élaboration d'un texte complet et abouti. Toutefois, la méthode employée par le Gouvernement et la majorité présidentielle lors du second passage de ce texte à l'Assemblée nationale n'est pas excusable. excusable. Le Sénat avait voté un certain nombre de dispositions visant à améliorer notre système de santé, pour reprendre la terminologie de l'intitulé de cette proposition de loi. Or, avec une méthode quasi binaire, vous avez alterné rétablissement de la version votée en première lecture par l'Assemblée nationale et suppression des articles additionnels votés par le Sénat.

À titre personnel, je me réjouis tout de même que la vaccination par les biologistes et les pharmaciens hospitaliers ait été conservée dans la version votée par l'Assemblée nationale. Cela étant, le cheminement de ces amendements est assez symptomatique de l'impréparation et des hésitations de l'exécutif face à cette crise sanitaire. L'amendement visant à permettre aux biologistes de vacciner a été voté en séance publique au Sénat. Par la suite, il a été supprimé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, avant de revoir le jour en séance publique avec une forme de bienveillance de la part du Gouvernement. Même si je suis satisfaite du résultat, ces péripéties m'interrogent sur la capacité du Gouvernement à déterminer un cap clair et précis et, surtout, à s'y tenir. Eh oui ! De la même manière, je m'interroge quant au cheminement de l'amendement tendant à permettre une prise de rendez-vous directement chez les orthophonistes. Cette disposition, votée par la Haute Assemblée, répondait à un principe de réalité- notre collègue vient de le rappeler. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait conservé cet apport de bon sens. Pourtant, le Gouvernement est revenu sur le consensus obtenu en modifiant cette disposition en séance publique. Madame la ministre, je regrette ce type de méthode, qui ne respecte pas le travail des commissions concernées. Les difficultés structurelles de notre système de santé ne sont en rien résolues : on reporte inlassablement ces sujets vers des textes futurs et hypothétiques, dont les titres sont vecteurs d'espoir et les contenus parfois créateurs de désespoir.

Vous l'aurez compris, cette méthode ne nous satisfait pas ; ce texte ne nous satisfait pas. Pis encore qu'une divergence idéologique profonde qui justifierait une opposition frontale de notre part, cette proposition de loi n'est tout simplement pas à la hauteur. Plus qu'un rendez-vous raté, c'est un rendez-vous manqué.

est à Mme la présidente de la commission, pour la motion. En application de l'article 44, alinéa 3, de notre règlement, la commission des affaires sociales a déposé sur ce texte une motion tendant à lui opposer la question préalable, afin de manifester l'opposition du Sénat à l'ensemble de ses dispositions. il ne s'agit pas pour la Haute Assemblée de rejeter le détail de toutes les mesures contenues dans la proposition de loi- certaines d'entre elles sont d'ailleurs le fruit de réflexions que nous avons conduites -, mais de prendre acte de l'incompatibilité des positions de nos deux assemblées et, ainsi, de l'inutilité de poursuivre plus avant nos débats. La discussion générale a montré en termes éloquents que les espoirs initialement soulevés par ce texte, gros de la belle unanimité sortie des accords du Ségur, ont été cruellement déçus par la modestie de ses dispositions. Je considère pour ma part que la nette aggravation de la situation sanitaire, dont nous venons de débattre devant le Gouvernement, oblige désormais à adapter nos discussions à la gravité des enjeux.

les organisations que nous avons déjà votées. Nous pensons également aux hôpitaux de proximité, qui représentent une réelle avancée pour la structuration des soins hospitaliers : ils répondent à la demande des acteurs de terrain, que vous-mêmes relayez régulièrement.

pour maintenir une activité. Il pourra désormais rappeler que le plafond réglementaire s'applique avec un contrôle par le comptable public et qu'il n'y a aucune dérogation possible. C'est un dispositif puissant, qui répond à un engagement fort. Enfin, s'agissant des compétences professionnelles, les deux chambres ont permis des avancées concrètes pour plusieurs professions. Je pense en aux sages-femmes, citées par Mme Doineau, qu'il s'agisse de la prescription d'arrêts de travail sans limitation de durée, de l'actualisation de la liste des médicaments dont la prescription leur est ouverte, de l'adressage par la sage-femme à un médecin spécialiste ou encore la déclaration d'une sage-femme référente. Je pense également aux masseurs-kinésithérapeutes et aux orthophonistes : le renouvellement de l'accès à ces professionnels dans l'année qui suit la prescription est rendu possible. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, cette proposition de loi comporte de nombreuses avancées

et les fondations. Le terme « contrat » est profondément mal employé. Il laisse entendre qu'une association pourrait exister sans respecter nos principes et lois communes. En outre, cette charte n'empêchera nullement un élu local d'islamo-clientélisme- elle pourrait même le couvrir. De même, elle n'aura aucune contrainte réelle sur les agissements d'une association séparatiste ou islamiste qui l'aurait signée en pratiquant une stratégie de, c'est-à-dire de dissimulation. Il existe déjà beaucoup trop de chartes non appliquées : n'en rajoutons pas ! Notre peuple n'a jamais vaincu ses ennemis en leur faisant signer une charte, mais en établissant un plan de guerre et de résistance Par ailleurs, cet amendement tend à renforcer la législation afin d'autoriser le retrait de subventions aux associations et aux fondations qui favorisent notamment le communautarisme islamiste ou qui sont inspirées par des idéologies de nature à troubler l'ordre et la paix publics en provoquant des tensions et divisions au sein de la communauté nationale,

qui aurait obtenu une subvention en usant d'un objet trompeur. Cette mesure financière punitive est bien plus dissuasive que le contrat d'engagement républicain prévu par cet article. devons en finir avec la dilapidation de l'argent public auprès d'associations qui participent au délitement de notre nation et nourrissent nos ennemis. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter mon amendement, qui se veut réaliste, réactif, pragmatique et efficace. Je le résumerai par ces quelques mots moins de chartes, plus de charters

retirerait toute référence aux principes républicains que nous soutenons aujourd'hui.

nous estimons que la charte des engagements réciproques constitue la réponse intelligente à la question posée. Nous sommes de fervents défenseurs des associations- Jean-Pierre Sueur a eu l'occasion de le rappeler hier soir. soir. Nous disons donc oui à la charte des engagements réciproques entre l'État, le mouvement associatif et les collectivités locales et non au contrat d'engagement républicain

Il n'y a aucune raison de limiter l'engagement à respecter les principes de la République aux seules associations, alors qu'elles concourent, au quotidien, à leur mise en oeuvre. Aussi Aussi proposons-nous d'étendre ce dispositif à l'ensemble des personnes morales sollicitant une subvention, un prêt ou une garantie de prêt auprès d'une autorité publique. Les entreprises qui bénéficient de subventions, de prêts ou de garanties de prêts publics devraient également s'engager à respecter ces principes. Il s'agit d'une mesure d'équité vis-à-vis des associations et des fondations, que celles-ci ont réclamée. Les associations sont déjà tenues à des obligations comptables et fiscales très lourdes par rapport aux sociétés de droit commun.

les principes républicains s'appliquent à tous les citoyens et, donc, à toutes les associations en vertu de la Constitution de la République française.

auxquels la France est attachée. Tel est l'objet de cet amendement. Il s'agit de nouveau d'un amendement de repli. Depuis une vingtaine d'années, les associations qui demandent une subvention à caractère public doivent souscrire à la charte des engagements réciproques, signée entre l'État, les associations d'élus et le mouvement associatif en 2001 rénovée en février 2014. Elle est ainsi jointe au formulaire Cerfa de demande de subvention. Cette charte porte déjà l'engagement de promouvoir et de faire respecter toutes les valeurs de la République, ainsi que d'ouvrir à tous les actions financées sans distinction d'origine, de religion ou de sexe. Tout manquement à ces principes peut conduire à la dénonciation de la subvention et à son reversement au Trésor public. L'intérêt de la mise en place d'un contrat d'engagement républicain pose donc légitimement question. En vertu des engagements liés à cette charte,

qui est donc susceptible d'être octroyée sous forme de mise à disposition de locaux. Le problème est que les élus ne savent souvent pas comment faire appliquer les règles existantes, ou ne le souhaitent pas pour des motifs divers. Il ne sert donc à rien de créer un contrat d'engagement républicain : il ne changera rien aux problèmes rencontrés par les élus ! Loin de constituer une solution miracle, il aura pour effet de stigmatiser une certaine catégorie d'administrés et d'obliger toutes les associations souhaitant obtenir une subvention publique à compléter leur objet pour coller aux termes de ce contrat. Nous préférons conférer une base légale à la charte des engagements réciproques.

il est spécifié que le décret précisant les modalités d'application de l'article fixera un seuil de montant de la subvention en deçà duquel l'adhésion à la charte ne sera pas requise. Il est inadmissible d'entamer la liberté d'association au point

Le contrat reste une faculté, mais inverse la logique d'obligation puisque ce n'est pas l'émetteur qui s'engage. Deuxièmement, en lien avec l'absence de négociation, ce contrat n'est aucunement plus protecteur que la charte des engagements réciproques signée entre l'État, les collectivités territoriales et les associations. cette dernière, qui a au moins le mérite d'exister et de faire l'objet d'un consensus, inscrit, elle aussi, la question des valeurs républicaines en son coeur. Troisièmement, la jurisprudence en matière de subventionnement des associations prévoit déjà largement l'obligation du respect des valeurs fondamentales. Ainsi, les collectivités publiques ne peuvent légalement subventionner que des activités présentant un intérêt public. Cette condition n'est pas satisfaite si l'action de l'association s'avère incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique ou des valeurs essentielles de la société. Les collectivités ont même le pouvoir de retirer une subvention en s'appuyant notamment sur des conventions d'objectifs et de moyens, bornées par la loi. Je concède que la commission du Sénat a légèrement amélioré le texte en définissant le contrat d'engagement républicain-

Pourtant, c'est leur mobilisation qui a abouti à l'adoption de la loi instaurant le droit au logement opposable. De même, que penser des associations qui, dans leur mode d'action, peuvent troubler l'ordre public- je pense notamment

dernier, « dans un texte principalement destiné à conforter la laïcité, il serait paradoxal que celle-ci ne soit pas explicitement incluse dans la charte d'engagement qui s'imposerait à toutes les associations percevant des subventions publiques À cet égard, on ne saurait objecter que des associations ayant une orientation religieuse ne pourraient respecter le principe de laïcité. Cette dernière vise, avec la séparation entre l'État et les cultes, à garantir le respect absolu de la liberté de conscience. On ne peut exonérer de ce respect une association signataire du contrat d'engagement républicain, quelle que soit la philosophie qui l'inspire. On peut même souhaiter qu'une association subventionnée par une autorité administrative,

S'il est légitime d'attendre des associations qu'elles s'abstiennent de commettre des infractions pénales, leur demander de s'engager de manière explicite sur des principes qui, rappelons-le, découlent de prérogatives de puissance publique, du maintien de l'ordre public en l'espèce, est tout de même déconcertant.

En outre, l'appréciation de la notion d'ordre public et les restrictions qui en découlent ne peuvent se faire que sous le strict contrôle du juge et du Conseil d'État. Les associations lanceuses d'alerte, les associations militantes de défense de l'environnement et de la condition animale, ainsi que les associations d'aide aux migrants seront mises en péril par l'établissement d'un tel contrat, dont les appréciations subjectives de menace à l'ordre public pourraient leur être opposées. Les associations sont des tiers essentiels à la vitalité de notre démocratie. Nous devons préserver leur liberté d'action et leur capacité de plaidoyer. La

avec les associations. Il en ressort qu'une « menace » peut être qualifiée préventivement à un trouble effectif à l'ordre public. Les termes « de nature à » nous semblent renforcer encore ce caractère hypothétique.

Le Gouvernement souhaite ajouter à l'article 1 de la Constitution que la République garantit la préservation de l'environnement et la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Ces principes existent déjà dans la Charte de l'environnement, ajouté au préambule de la Constitution en 2005. Ces principes nous obligent collectivement, dans leur ensemble. Conforter l'un ou l'autre des principes, en oubliant les autres, n'est que le reflet d'obsessions. Les six heures de débat sur le voile n'ont fait qu'affermir une vision stigmatisante de la République. Si nous sommes opposés au principe même du contrat d'engagement républicain, nous souhaitons qu'il soit tout de même enrichi. Nous proposons d'inscrire dans les obligations des signataires du contrat la nécessité de respecter la Charte de l'environnement. Les dérèglements du climat et l'effondrement de la biodiversité vont aussi fragiliser et mettre en tension notre République. La préservation de nos biens communs doit devenir un principe républicain unanimement partagé. Si aucun euro d'argent public ne doit aller à des structures qui remettent en cause la laïcité, aucun euro d'argent public ne doit non plus aller à celles et ceux qui s'attaquent à des espèces protégées ou qui saccagent notre environnement.

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère propre de l'enseignement privé, les associations qui ont une aspiration spirituelle et qui s'expriment publiquement à ce titre doivent pouvoir continuer à le faire.

est à M. Julien Bargeton. Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour les fondations d'informer leurs membres de leur engagement à respecter les principes républicains résultant du contrat d'engagement républicain, introduite lors de l'examen du texte en commission. En effet, les fondations correspondant à un rassemblement de biens, elles ne possèdent pas de « membres » à proprement parler, contrairement aux associations, qui, elles, constituent un rassemblement de personnes. La coordination à laquelle il a été procédé ne semble donc pas opportune. L'amendement

Pour autant, effectivement, la République est laïque. C'est pourquoi nous proposons, pour que la laïcité apparaisse malgré tout dans ce texte, d'imposer aux associations de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République,

J'en viens à la dernière série d'amendements. L'amendement n° 307 de M. Dossus tend à intégrer dans le contrat d'engagement républicain l'obligation pour les associations d'oeuvrer pour la protection de l'environnement et, surtout, de s'assurer du respect du principe de précaution.

et les hommes. Si c'est stigmatisant de dire à des associations « d'accord, on vous donne des subventions, mais on attend de vous que vous respectiez l'égalité entre les femmes et les hommes et les grands principes de la laïcité », alors les mots n'ont plus de valeur et rien n'est stigmatisant

enceintes. L'amendement n° 307 tend à prévoir que les associations bénéficiant de subventions doivent oeuvrer pour la préservation et l'amélioration de l'environnement et s'assurer du respect du principe de précaution défini dans la Charte de l'environnement. Nous sommes bien évidemment favorables à tous ces principes.

Je vous le dis très simplement. Le monde associatif représente 1,5 million d'associations, 13 millions de bénévoles et 1,8 million de salariés. Ces salariés sont d'ailleurs souvent qualifiés, occupent des emplois pérennes et non délocalisables. C'est une force et une richesse pour notre pays.

enrichie par la charte des engagements réciproques, durement négociée avec le monde associatif en 2001, puis enrichie en 2014. Je ne

J'ajouterai toutefois une chose qui me paraît importante. Je veux bien laisser passer cet article 6, mais je ne veux pas en être dupe. Je considère que cet article est une illusion, un coup d'épée dans l'eau. ! Il contribue à me faire penser que l'ensemble de ce texte est un tigre de papier. Tout le monde signera le contrat d'engagement républicain. Je

et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, au sens de l'article 2 de la Constitution. Toutes les associations de France doivent s'abstenir de remettre en cause le caractère laïque de la République. Toutes les associations de France doivent s'abstenir de toute action de nature à constituer une menace pour l'ordre public. public. Si seules celles qui signent le contrat d'engagement étaient assujetties à ces obligations, qui s'imposent à tout citoyen français à vrai dire, alors la République serait sens dessus dessous. Ce serait très grave ! Je ne voudrais pas que notre texte puisse avoir une implication si dangereuse. Alors, oui, laissons passer cet article 6. Donnons sa chance au Gouvernement. Il va arrêter la déferlante de l'islamisme radical grâce aux employés de bureau des préfectures qui vérifieront le contrat d'engagement. Les Français peuvent être rassurés, moi pas

explication de vote. Après le plaidoyer de notre collègue Philippe Bas, je m'en voudrais d'en rajouter. Je partage bien évidemment en tout point ce qui vient d'être dit, et j'ai les mêmes inquiétudes sur l'intérêt de cet article.

L'article 6 parle de la vie associative, qui est aussi une richesse morale, intellectuelle.